La séance est ouverte.

Monsieur le Premier ministre, au nom du Sénat tout entier, je tiens de nouveau à vous féliciter pour votre nomination et vous souhaiter la bienvenue au sein de notre assemblée dans vos nouvelles fonctions. Depuis le début de la législature, votre prédécesseure, Mme Élisabeth Borne, a témoigné, lors de nos séances de questions d’actualité, d’une présence constante à laquelle nous avons été particulièrement sensibles et que je tiens une nouvelle fois à saluer. Je souhaite également la bienvenue aux membres du Gouvernement, avec une attention particulière pour la ministre chargée des relations avec le Parlement, Mme Marie Lebec. Monsieur le Premier ministre, mesdames, messieurs les ministres, le Sénat est le reflet de nos territoires, dans leur diversité. Sur ses travées siègent des élus expérimentés, qui sont à l’écoute de nos concitoyens et de nos collectivités territoriales.

dans votre nouveau monde, un monde fait pour les riches, un monde d’oppression pour les salariés, un monde qui exclut au lieu de rassembler. Cette politique engendre une crise démocratique profonde. D’ailleurs, le Président de la République n’a toujours pas de majorité absolue à l’Assemblée nationale. Cette question n’est ni politicienne ni secondaire : c’est le socle du fonctionnement de nos institutions. Vous ne pouvez plus faire jouer l’autoritarisme, en abusant du 49.3 comme en 2023. Continuerez vous d’user de cet article de la Constitution ou vous engagez

C’est fondamental, car si le Gouvernement se mue en un cabinet d’exécutants, sans vote de confiance du Parlement, c’est l’édifice institutionnel qui s’effondre. Emmanuel Macron prend tout en main,

a soif de justice. Votre mandat doit être soumis au vote des représentants du peuple ; à défaut, vous ne serez qu’illusion. Je vous repose donc la question, monsieur le Premier ministre : allez vous demander la confiance

J’ai eu l’occasion de le dire, je ferai ma déclaration de politique générale à l’Assemblée nationale le 30 janvier prochain, parce que je souhaite, d’ici là,

pour valoriser le travail des classes moyennes, qui sont toujours au rendez vous de leurs responsabilités et qui attendent que l’on agisse pour elles, pour réarmer nos services publics, notamment l’école et la santé pour assurer la sécurité en tout lieu sur le territoire et pour agir en faveur de la transition écologique. Voilà les préoccupations des Français ! Je peux

Il n’a en revanche pas ou peu évoqué un sujet qui nous paraît pourtant important : la situation de nos finances publiques. Nous atteignons un record de dette, qui nous place sur le podium européen des pays les plus endettés, notre charge de la dette va bondir de 50 % d’ici à 2027 et notre déficit sera le deuxième plus important de la zone euro. Plusieurs annonces du Président vont même encore aggraver cette situation : généralisation du service national universel (SNU), qui pourrait coûter plus de 3 milliards d’euros par an, et baisse de 2 milliards d’euros des impôts. Mes questions sont donc très simples. À combien chiffrez vous les annonces du Président de la République ? Comment comptez vous les financer ? Quelles sont les intentions réelles du Gouvernement en termes de maîtrise des finances publiques, sujet souvent évoqué, mais jamais réalisé ?

mes meilleurs vœux. Monsieur Maurey, nous nous connaissons bien – nous avons été élus du même territoire pendant une quinzaine d’années – et vous savez que j’ai l’habitude de faire les choses en temps et en heure. À partir de 2017, avec les gouvernements précédents, nous avons rétabli nos finances publiques. J’avais dit que nous reviendrions sous les 3 % de déficit et que nous sortirions de la procédure pour déficit public excessif : j’ai tenu parole.

Vous avez appelé à une protection des plus modestes face à la crise inflationniste et à la flambée des prix du gaz et de l’électricité : nous l’avons fait. Désormais, nous revenons à la normale et sortons d’une situation exceptionnelle. Je partage totalement votre ambition et je tiendrai parole : nous devons rétablir nos finances publiques, accélérer le désendettement du pays et réduire nos déficits, en tenant la première marche de 2024 – 4,4 % de déficit – et en accélérant ensuite. Je crois avoir dit les choses très clairement il y a quelques semaines : en matière de finances publiques, le plus dur est devant nous ! Pour les Français ! Nous allons devoir prendre des décisions fortes et courageuses pour rétablir nos finances publiques.

et au Président de la République des décisions fortes et courageuses. Je n’ai aucun doute, monsieur le sénateur, que vous les soutiendrez. La parole Maurey, pour la réplique. Monsieur le ministre, vous n’avez pas tout à fait répondu à mes questions, mais je ne m’attendais pas à autre chose. Je voudrais simplement dire qu’il me paraît difficile, en matière de finances publiques, de pratiquer le « en même temps On ne peut parler d’indépendance financière, comme l’a fait le Président de la République, et continuer de dépenser et de s’endetter chaque jour davantage. Vous avez dit récemment qu’il faudrait faire 12 milliards d’euros Le moins que l’on puisse dire, c’est que les mesures évoquées par le Président de la République ou celles que le Premier ministre a annoncées, soit 32 milliards d’euros supplémentaires pour la santé, ne vont pas dans le bon sens. De toute évidence, la valse des milliards continue et la loi de programmation des finances publiques, à peine votée, semble déjà caduque… Je voudrais juste rappeler que le Sénat, lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2024, a proposé 7 milliards d’euros d’économies et 2 milliards d’euros de recettes supplémentaires.

La situation à Gaza, elle, ne peut plus attendre. En cent jours, 1 % des Gazaouis ont été tués, soit un taux de mortalité quotidien supérieur à celui de n’importe quel conflit armé du XXI siècle, sans compter les personnes ensevelies et blessées, et 85 % ont été déplacés.

que le monde fasse quelque chose. » Nous savons ! Vous savez ! La France a la responsabilité et l’obligation, en tant qu’État partie aux conventions internationales, de protéger et d’agir pour mettre un terme aux crimes de guerre, aux crimes contre l’humanité, voire au génocide en cours à Gaza comme partout dans le monde, et sans double standard En Ukraine comme en Palestine se jouent la défense des principes fondamentaux du droit international et l’avenir de l’Europe. Le massacre de civils doit cesser. Quelles mesures comptez vous prendre pour faire respecter le droit international et ses résolutions ? Vous engagez vous à appuyer et à faire appliquer les mesures conservatoires demandées à la CIJ ? Vous engagez vous

Comptez vous décider un embargo sur les ventes d’armes à Israël ? Enfin, monsieur le ministre, quand comptez vous reconnaître l’État palestinien, comme cela a été voté par notre Parlement, et soutenir l’Espagne dans cette demande auprès de l’Union européenne ?

de façon dramatique. Dans cette guerre, l’action de la France se fonde sur trois volets, qui ont été fixés par le Président de la République. Le volet sécuritaire, tout d’abord. La lutte contre le terrorisme passe notamment par l’adoption prochaine d’un régime de sanctions européennes

et cessez le feu durable – il est nécessaire pour permettre l’acheminement de l’aide. La France a d’ores et déjà déployé 1 000 tonnes de nourriture et d’équipements et 100 millions d’euros pour les populations palestiniennes.

Ma question s’adresse à M. le Premier ministre. À l’occasion des discussions sur le projet de loi Immigration, une partie du débat s’est nouée autour de l’aide médicale de l’État

Dans le contexte de la guerre entre Israël et le Hamas, la tension est montée en mer Rouge ces dernières semaines avec des attaques des Houthis visant le trafic maritime, en solidarité avec la bande de Gaza. Cette voie stratégique, qui relie la Méditerranée à l’océan Indien, est cruciale pour le commerce mondial, quelque 20 000 navires la traversant chaque année. Depuis mi octobre, cette route commerciale est menacée par les Houthis, des rebelles yéménites membres d’une organisation soutenue par l’Iran voulant interdire le passage aux navires des pays qu’ils estiment être proches d’Israël. Cette milice yéménite a rejoint la coalition informelle appelée Axe de la résistance, qui réunit notamment l’Iran, le Hamas et le Hezbollah contre l’État d’Israël. Cette coalition fait planer le spectre d’un conflit généralisé. La France fait partie de la coalition internationale assurant la sécurité en mer Rouge. En décembre dernier, la frégate, en mission en mer Rouge, patrouillant dans la zone, a abattu en légitime défense des drones se dirigeant vers elle. Ces attaques houthies dissuadent les navires commerciaux d’emprunter la mer Rouge. Ils se détournent du canal de Suez, optant pour le cap de Bonne Espérance. Cette route alternative allonge considérablement leur trajet, ce qui entraîne une hausse du tarif des transports. Ces attaques menacent la libre circulation du commerce et violent le droit international. La liberté de navigation en mer Rouge est d’une importance cruciale pour les intérêts de la France, ne serait ce que pour assurer les liaisons maritimes avec ses territoires de l’océan Indien, Mayotte et La Réunion. Cette situation aggrave l’inflation sur les produits importés dans ces territoires. La crise en mer Rouge ne constitue pas seulement un danger sur le plan sécuritaire, c’est aussi un danger commercial avec des répercussions qui entraînent une pression inflationniste sur la France et l’Europe et qui pénalisent l’économie mondiale. Monsieur le ministre, face à cette double menace sécuritaire et commerciale en mer Rouge, quelles mesures envisagez vous pour protéger les intérêts commerciaux et économiques de la France ?

les Houthis menacent la sécurité maritime et le commerce international en mer Rouge. Ces attaques sont une atteinte à nos intérêts nationaux et aux intérêts européens. Un navire de la CMA CGM et la frégate ont d’ailleurs été directement ciblés. Plusieurs compagnies maritimes, vous l’avez dit, sont contraintes de contourner cette zone. Ces attaques sont aussi une violation évidente du droit international. La résolution adoptée le 10 janvier dernier par le Conseil de sécurité des Nations unies les condamne et rappelle le droit des États à se défendre.

Dans ce contexte, les États Unis ont fait le choix d’une opération militaire sur les territoires contrôlés par les Houthis. La France n’a pas souhaité y prendre part. À ce stade, nous nous contentons de mener une action en mer en totale autonomie, mais en coordination avec nos alliés. Nous étudions aussi les moyens de renforcer la présence européenne en mer Rouge.

Il faut maintenant tenir cette promesse ! La situation est devenue critique. Les crimes de guerre du boucher du Kremlin infligent chaque jour un atroce supplice à la population civile d’Ukraine. Les Ukrainiens, qui ont brillamment contre attaqué à Kharkiv et Kherson en 2022, sont aujourd’hui en position de faiblesse, parce que, depuis le début, le soutien des démocraties peut se résumer par une formule : trop peu, trop tard ! Si nous avions livré à temps les chars, les missiles, les batteries anti aériennes, l’armée russe n’aurait pu reconstituer ses défenses et faire échouer la contre offensive de 2023. Nous sommes en train de renouveler cette erreur. Depuis des mois, Zelensky attend 60 milliards de dollars de Washington, bloqués par les Trumpistes au Congrès, et 50 milliards d’euros de l’Europe, paralysée par ses cinquièmes colonnes – Orbán le collabo en Hongrie, Le Pen et Mélenchon, les chiens chiens à leur Poutine en France, et tant d’autres ailleurs. Nos tergiversations mettent l’Ukraine en grand danger – je pèse mes mots. Une défaite serait celle de l’Europe tout entière, un formidable stimulant pour la Chine face à Taïwan, pour le docteur Folamour de Corée du Nord, pour les mollahs iraniens tueurs de femmes au Moyen Orient. Il serait impensable que le prochain Conseil européen du 1 février ne déjoue pas les manœuvres d’Orbán le corrompu et ne débloque pas la totalité de l’aide promise à l’Ukraine. Je vous demande aujourd’hui

En ce début de mandat, vous vous dites sans doute, monsieur le Premier ministre, que vous serez jugé sur vos résultats dans notre pays, et c’est exact. Mais à l’échelle de l’Histoire, votre gouvernement et tous les gouvernements d’Europe seront jugés à l’aune de la victoire ou de la défaite des démocraties en Ukraine face à l’internationale reconstituée des dictateurs.

voilà près de deux ans, en dépit de toutes les règles de droit international et de tous ses engagements, la Russie a agressé l’Ukraine. C’est une attaque cynique et meurtrière, avec des frappes aériennes répétées, qui visent délibérément les civils. Ce qui est en jeu dans ce conflit – je vous remercie de l’avoir rappelé aussi clairement –, c’est la liberté, la démocratie et l’avenir de notre continent. La Russie espère que l’Ukraine cédera et que ses soutiens se lasseront. Je le dis de manière très claire, en tant que chef du Gouvernement, comme le Président de la République l’a rappelé hier : la Russie se trompe. l’a rappelé hier : la Russie se trompe. Nous ne faiblirons pas et nous ne faiblirons jamais. Notre détermination est intacte, je le réaffirme ici devant vous. Le ministre de l’Europe et des affaires étrangères s’est rendu à Kiev pour son premier déplacement après sa nomination. Permettez moi, pour la première fois en tant que Premier ministre, au nom du Gouvernement, et en votre nom à tous, j’en suis sûr, de dire mon admiration pour le peuple ukrainien et de saluer son courage exceptionnel. Monsieur le président Malhuret, vous avez évoqué notre soutien à l’Ukraine, lequel, je le disais à l’instant, ne faiblira pas. Le Président de la République a annoncé hier la livraison de nouveaux missiles de longue portée et de centaines de bombes. Ce sont des armements attendus par les Ukrainiens et qui seront déterminants sur le terrain. En parallèle, nous continuons à former des militaires ukrainiens, comme nous le faisons depuis le début du conflit pour répondre à leurs besoins. Nous poursuivrons donc notre soutien militaire, en concertation avec nos partenaires. J’ajoute que notre soutien humanitaire continue lui aussi, pour répondre aux besoins les plus immédiats du peuple ukrainien, notamment en matière d’éducation et de santé. la mobilisation de tous les acteurs est essentielle. Je pense évidemment à l’État, aux collectivités locales, dont je veux saluer l’engagement remarquable. Nombre d’entre elles interviennent en solidarité avec les Ukrainiens. Je pense aussi aux acteurs privés, engagés en soutien de l’économie ukrainienne, dans la perspective de la reconstruction. Notre soutien de long terme à l’Ukraine civile comme militaire sera inscrit dans l’accord bilatéral de sécurité que que le Président de la République signera avec le président Zelensky, lors de son déplacement à Kiev en février prochain. Ce soutien de la France, le Président de la République aura l’occasion de le réaffirmer vendredi, à Cherbourg, en adressant ses vœux à nos armées. J’ajoute, comme vous l’avez rappelé, que la France porte également la mobilisation en faveur de l’Ukraine à l’échelon européen. Nous sommes déterminés à obtenir un accord sur la Facilité pour l’Ukraine au Conseil européen extraordinaire du 1 février prochain. Concrètement, cette facilité doit permettre à l’Ukraine de faire face à ses besoins de financement immédiats et de mener les investissements essentiels pour se reconstruire et se moderniser. L’Union européenne est également déterminée à poursuivre son soutien militaire à l’Ukraine. Le Conseil européen de décembre dernier a ainsi demandé que s’intensifient les travaux sur la réforme de la Facilité européenne pour la paix (FEP). En s’en prenant à l’Ukraine, la Russie a attaqué nos valeurs. La Russie a remis en cause la démocratie et la liberté. Nous nous tiendrons aux côtés de l’Ukraine et du peuple ukrainien. Nous nous tiendrons toujours aux côtés de nos valeurs, c’est l’une de nos priorités. La parole est à Mme Nathalie

interrogeait le ministre de l’agriculture de l’époque, Didier Guillaume, sur la manière dont il comptait venir en aide aux ostréiculteurs, alors durement touchés par des pollutions de l’eau de mer au norovirus, lors des fêtes de fin d’année de 2019. Mme Élisabeth Borne, alors ministre de la transition écologique, rappelait que, dans le cadre du onzième programme d’intervention des agences de l’eau, quelque 3,6 milliards d’euros d’aides devaient être accordés au titre du traitement des eaux usées. Comment et où ces fonds ont ils été employés ? Force est de constater que les mêmes causes ont produit les mêmes effets. En témoigne l’interdiction de la vente d’huîtres du bassin d’Arcachon prise par arrêté préfectoral le 27 décembre dernier, en raison de la contamination de la production au Le préfet a réuni autour de lui les collectivités et les établissements publics compétents dans la gestion des eaux usées et des eaux pluviales sur le bassin versant. Il a promis d’accélérer les programmes d’investissement pour apporter des réponses à moyen et long termes.

La fermeture pour vingt huit jours de la totalité de la zone de production du bassin d’Arcachon a entraîné 5 millions d’euros de pertes sèches et fait craindre de perdre la confiance des consommateurs.

réseaux d’eau pluviale, qui étaient saturés, ont conduit à la propagation du norovirus, qui produit des infections humaines de type gastroentérite aiguë. Une telle situation a justifié les mesures de protection prises par la direction générale de l’alimentation. Les interdictions temporaires sont destinées à protéger

à la suite d’un épisode de filtration dans des eaux saines, le préjudice économique et le préjudice d’image, c’est à dire le préjudice médiatique, sont importants. Puisque les producteurs ne sont en rien responsables, la possibilité de mobiliser des mesures de soutien, cela a été dit

Monsieur le président, monsieur le Premier ministre, dans un exercice assumé d’autosatisfaction, le président Macron m’a hier rassuré. Notre pays va bien, l’ascenseur social fonctionne et nos services publics ont les moyens de remplir leurs missions J’ai sans doute été distrait, car, pour moi, la réalité est tout autre. Dans ma réalité, l’école publique est fragilisée par des professeurs non remplacés et désabusés. L’hôpital public s’effondre. J’ai en tête l’exemple tristement emblématique de la maternité Jeanne de Flandre, à Lille, qui transfère une partie de ses patientes et de leurs bébés en Belgique. Dans ma réalité, la France compte désormais près de 5 millions de pauvres et la classe moyenne a de plus en plus de mal à joindre les deux bouts. Le déclassement social frappe de plus en plus nos concitoyens. Dans ma réalité, le logement traverse une crise d’une ampleur inédite depuis trente ans, sans que nous disposions, à ce stade, d’un ministre de plein exercice. Monsieur le Premier ministre, il faut ouvrir les yeux. Tel est l’état de la France, dont vous êtes comptable. Les propos du Président de la République traduisent sa déconnexion avec le quotidien des Français. Pour lui, c’est la moralisation et l’ordre pour les citoyens, la dérégulation et le désordre pour les intérêts financiers. Ce n’est pas d’optimisme dont il a fait preuve hier soir : il cultive une amnésie politicienne pour conserver le mauvais cap qu’il a fixé voilà bientôt sept ans. Quant aux Français, ils n’ont rien oublié : ni l’injuste réforme des retraites, ni la stigmatisation des chômeurs, ni la xénophobie rampante de la loi Immigration. Monsieur le Premier ministre, aurez vous la lucidité de poser ce constat ? Aurez vous l’audace d’en tirer toutes les conséquences ?

ou sourd aux difficultés que traversent les Français et à la situation du pays ? La réponse est non. Je crois l’avoir dit dès ma prise de fonction à Matignon, lors de la passation de pouvoir : je suis lucide sur les difficultés, les angoisses, les inquiétudes, les doutes et les colères de nombreux Français.

qui ont toujours le sentiment d’avoir un peu plus de ce qu’il faut pour être accompagnés par la solidarité nationale et un peu moins de ce qu’il faut pour s’en sortir tout seuls, attendent beaucoup de nous.

France un pays moteur en matière de transition écologique. J’entends les critiques et les questions qui sont posées, mais j’attends que l’on me montre un pays de l’Union européenne qui s’engage autant que nous, un pays ayant réussi à réduire de 4 % ses émissions de gaz à effet de serre, comme nous l’avons fait l’an dernier ! Quel pays a réussi à faire la même chose dans l’Union européenne ?

pour la réplique. Monsieur le Premier ministre, je ne doute pas de votre sincérité. Simplement, je vous le dis comme je le pense : changer de premier violon ne change pas la partition.

de la jeunesse, des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques. J’espère, madame, n’avoir oublié aucune de vos fonctions…

À la lumière de votre large portefeuille, comment comptez vous concilier de manière efficace et permanente la bataille de la refondation de l’école et, en même temps, le défi de l’organisation des Jeux de Paris ? Dans cette « mère des batailles », quelle image du professeur entendez vous porter dans la société ? Quelle est votre vision de son rôle, de sa place, de son autorité ? Dans cette « mère des batailles », quel rôle et quelle place entendez vous donner à l’enseignement privé, sous contrat et hors contrat ? sports et des jeux Olympiques et Paralympiques. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, monsieur le sénateur Max Brisson, en réunissant les champs de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports dans notre contexte olympique et paralympique, vous n’avez rien oublié Le Président de la République et le Premier ministre m’ont confié un continuum de responsabilités aux synergies nombreuses. Au cœur de ce continuum, il y a une ambition, à savoir le réarmement civique de notre jeunesse et il y a un trésor, c’est l’école. Pour la servir, je m’appuierai sur trois piliers. D’abord, il convient de restaurer l’exigence, au travers du choc des savoirs impulsé par Gabriel Attal, et de réaffirmer l’autorité de nos professeurs sur la vie de classe, leurs enseignements, les décisions de redoublement et les notations. Ensuite, il faut renforcer l’attractivité des métiers de l’enseignement, en réinventant la formation initiale des enseignants, en repensant leur formation continue, en continuant d’améliorer l’organisation et les remplacements de courte durée, en poursuivant les réformes engagées pour la revalorisation des carrières et des conditions de travail des enseignants et d’autres catégories de personnel, comme les infirmières scolaires, les assistants sociaux et les ! Enfin, il est nécessaire, plus que jamais, dans la France des jeux Olympiques et Paralympiques, de construire une école de l’épanouissement républicain, où la peur et le harcèlement n’ont plus leur place, une école dans laquelle tous les élèves s’approprient les valeurs de la République, avec l’instruction civique, le respect de la laïcité

pour la réplique. Madame la ministre, drôle de zigzag que le Président de la République fait subir à notre école ! Jean Michel Blanquer parlait laïcité, autorité et confiance, avant de constater, impuissant, malgré une avalanche de circulaires, la dégringolade de notre école. Pap Ndiaye passait par dessus bord les principes chers à son prédécesseur. Sous couvert de mixité sociale, il a sapé les derniers espaces d’excellence de notre école. Enfin, Gabriel Attal, pendant cinq mois et vingt jours, nous a offert une ode une ode quotidienne à l’école, dont nous attendons toujours la traduction en actes. Au lieu de zigzag, ne serait il pas temps de fixer un cap et de s’y tenir dans la durée, avec, pour valeurs cardinales, la liberté,

La parole est à Mme Audrey Bélim, pour le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain. et Républicain. Monsieur le Premier ministre, La Réunion a connu pour la première fois depuis trente ans le passage de l’œil d’un cyclone. Je profite de ce moment pour exprimer ma solidarité aux Mauriciens, également durement À l’heure où nous parlons, le bilan humain fait état de quatre décès. Sur le plan matériel, de nombreux Réunionnais sont sinistrés. Les récoltes des agriculteurs ont été fortement atteintes par le cyclone. Je salue l’action des élus locaux, qui ont ouvert dans des délais contraints 158 centres d’hébergement d’urgence pour les populations les plus fragiles, mais aussi celle du préfet et du Gouvernement. Vendredi devrait être annoncée la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle, demandée par l’Association des maires du département de La Réunion, que j’ai soutenue. Pour l’instant, La Réunion a tenu, mais Belal n’est qu’un avertissement de plus. La prévention des risques et la préparation face aux crises doivent être renforcées. À court terme se pose la question de l’accompagnement des collectivités. Par exemple, à Saint Denis, les dépenses post cyclones s’élèvent à 6 millions d’euros, et ce sans les travaux sur le bâti. À moyen terme se pose la question de la résilience de notre territoire. De nombreux Réunionnais n’ont plus accès à l’électricité ni à l’eau. Les budgets liés aux réseaux de distribution d’électricité sont ils à la hauteur des besoins ? Comment se fait il que les fils électriques ne soient pas enterrés, alors que La Réunion est une terre de cyclones ? Ce n’est pas une surprise, ce n’est pas imprévisible ! Une succession de cellules de crise ne pourra pas faire une politique. Se pose aussi la question de notre lutte contre le dérèglement climatique. Nous l’avons vu dans le Pas de Calais, nous le voyons aujourd’hui à La Réunion, les tempêtes et cyclones se multiplieront et s’aggraveront. Qu’allez vous faire pour accélérer en matière de transition énergétique, alors même que le ministère de plein exercice a été supprimé ? La question n’est donc pas de savoir ce qui a été fait, mais bien ce que vous allez faire !

par ce cyclone. Permettez moi de répondre très rapidement, mais avec précision, aux éléments importants que vous avez évoqués. L’alerte rouge a en effet été levée par le préfet hier à treize heures, heure locale. Les actions de reconnaissance se poursuivent et le déblaiement des voiries a débuté. Les coupures d’électricité, d’eau et de réseaux téléphoniques fixes comme mobiles ont été importantes, mais sont en cours de réparation. Les principaux réseaux routiers ont été rouverts à la circulation. Seuls les réseaux secondaires et la voie d’accès à Cilaos à Cilaos doivent encore faire l’objet de travaux de déblaiement. Sur le plan humain, nous déplorons quatre victimes. Le Président de la République a décidé l’engagement de moyens nationaux.

catastrophe naturelle, dont la commission devrait se réunir dès demain, madame la sénatrice. Avec le concours du préfet, l’ensemble des dispositifs d’appui aux populations exploitantes du monde agricole ou industriel

Ce crash de la natalité est destructeur pour notre économie et notre système social. Il constitue une menace existentielle pour notre pays, puisque le renouvellement des générations n’est plus assuré. Le recours à une immigration massive pour compenser ce déficit de naissances serait une très grave erreur. Cela risquerait de détruire la cohésion nationale. Le nombre d’enfants désirés par les familles reste largement supérieur aux naissances. la responsabilité du Gouvernement est immense. Que s’est il passé ces dernières années ? Le quotient familial a été rogné, les allocations ont été rabotées, les coûts de garde d’enfant ont augmenté, la prestation d’accueil du jeune enfant a diminué… et j’en passe

Des mesures ont d’ores et déjà été annoncées et mises en œuvre en 2023 : allongement du congé de paternité à vingt cinq jours, mise en place de l’entretien prénatal et postnatal précoce, investissement massif dans la recherche contre l’infertilité dans le cadre de France Relance.

Nous allons également accélérer la lutte contre la pénurie de professionnels de la petite enfance et renforcer l’attractivité des métiers. Tel est l’enjeu des revalorisations salariales annoncées, que nous allons mettre en œuvre en lien avec les branches et les communes. Enfin, le Président de la République a annoncé hier la mise en place d’un nouveau congé de naissance. Plus court, mieux rémunéré que le congé parental actuel, il permettra d’augmenter le temps de présence auprès des enfants sur les 1 000 premiers jours de la vie sans pénaliser les ménages

arrêtez de dépenser de l’argent public à coups de chèques et de subventions bidon, mais investissez pour la petite enfance et le pouvoir d’achat, soutenez financièrement et fiscalement toutes les familles, faites coexister congé parental court bien rémunéré et congé long moins rémunéré, soutenez la création de places de crèche et redonnez un ministère à la famille ! Ce sont les familles d’aujourd’hui qui préparent la France de demain. Il faut leur redonner espoir et confiance. Agissez vite

Monsieur le président, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, au matin de Noël, puis au matin du Nouvel An, Gabriel Bremond, maire d’Eclans Nenon, dans le Jura, découvre des tags partout dans le village et sur les murs de sa mairie

Gabriel Bremond est un maire sans histoires, apprécié de ses administrés. Il est solide. Il a déposé plainte et il fait face. Mais comment ? Les témoignages de sympathie de ses administrés lui apportent un réconfort salutaire, comme ceux des maires de toute la France, qui témoignent de la solidarité des membres de cette grande famille républicaine qu’il a choisi de servir et qui n’en finit pas d’être maltraitée 2 600 agressions l’an passé, 50 % de plus qu’il y a deux ans ! Malgré les indignations, malgré les textes votés, la dérive est implacable, insupportable. Monsieur le Premier ministre, vous avez déclaré, à Dijon, le week end dernier : « Nous sommes un gouvernement qui va continuer d’agir contre les discriminations, contre l’homophobie et en faveur des droits de tous. voyez vous ? – ces attaques démontrent que leurs auteurs n’ont ni peur des forces de l’ordre ni peur de la justice ! Notre République ne sait pas protéger ses maires. Monsieur le Premier ministre, qu’allez vous changer pour qu’ils soient respectés ?

Vous le savez, madame la sénatrice, dès mon arrivée à la Chancellerie, j’ai pris un certain nombre de circulaires claires pour demander expressément à tous les procureurs de notre pays une réponse systématique, une réponse ferme, une réponse rapide.

magistrats, greffiers, contractuels devenus attachés de justice. À Besançon, dans une cour d’appel dont je sais, madame la sénatrice, qu’elle vous est chère, cinquante huit de ces personnels vont arriver.

À gravité égale, pour des faits de violences, le taux de prononcé d’un emprisonnement ferme est de 51 % lorsque la victime est un élu, de 25 % lorsque la victime n’est pas un élu. Le taux de défèrement est cinq fois plus élevé, le d’un mandat de dépôt quatre fois plus élevé, lorsque la victime est un élu. Soyez assurée, Madame la sénatrice, Mesdames, Messieurs les sénateurs, que le combat continue et que notre engagement dans la défense des élus est

énergie des logements, notée de A à G, qui définit leur valeur et les autorise ou non à être loués, repose en réalité sur des calculs purement théoriques et sur une modélisation très approximative. Ainsi, le fameux « diagnostic de performance énergétique », ou DPE, transformé en quête du Graal climatique, pour lequel l’État investit des milliards d’euros, ne reflète pas la consommation réelle des logements ni les gains énergétiques Or c’est bien ce même DPE qui aggrave aujourd’hui une crise du logement sans précédent, notamment pour les locataires et propriétaires les plus modestes. Depuis le 1 janvier 2023, tous les logements classés G+ sont interdits à la location, et cette décision repose sur un algorithme biaisé. Que dites vous, monsieur le ministre, aux propriétaires et aux locataires qui en font d’ores et déjà les frais ? Si l’on persiste dans les échéances annoncées, 11 millions de logements classés F et G vont être interdits à la location dans les dix années à venir, sans véritable raison. Une fois de plus, cette machine à exclure retombera sur les maires, eux mêmes dépassés par la pénurie de logements et par les contraintes liées à la construction. Monsieur le ministre, qu’allez vous faire pour supprimer et remplacer cet outil défaillant, qui paralyse le secteur du logement ?

la réplique. Monsieur le ministre, ce n’est pas la première fois que l’on fonde une politique majeure sur des modélisations un peu fumeuses… Les Français perdent une nouvelle fois confiance dans cet État qui s’appuie sur un dispositif qui n’est bienveillant ni pour eux ni pour la planète.

La parole est à Mme Colombe Brossel, pour le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

Parlons de l’école de la République, l’école publique, laïque, gratuite et obligatoire. Cette école, c’est celle qui scolarise 80 % des élèves de ce pays, d’où qu’ils viennent. C’est vers elle C’est vers elle que votre énergie devrait être tournée, afin de garantir la réussite de tous, élèves comme personnel, car les défis sont immenses et vous êtes au pouvoir depuis plus de six ans. Vous avez, de fait, posé la question

Madame la ministre, quels moyens allez vous enfin donner à l’école publique pour la renforcer ? vraiment que l’on ne doit pas opposer l’école publique et l’école privée. C’est une autocritique ! Depuis la loi Debré du 31 décembre 1959, adoptée sous la présidence du général de Gaulle, qui établit la liberté d’enseignement dans notre pays, celui ci vit et vit bien avec des écoles publiques et avec des écoles privées.

et recrutés avec les mêmes exigences de qualification que dans le public. La moitié des familles ont eu recours au moins une fois à l’enseignement privé pour au moins un de leurs enfants

incapable de répondre à la question simple que je vous ai posée. Vous vous êtes mise toute seule dans une situation faite de polémiques et de mensonges. L’impuissance que vous projetez aujourd’hui est délétère pour l’école, alors que les enfants, les enseignants, l’ensemble des personnels, les parents, ont besoin de force

La parole est à M. Jean François Rapin, pour le groupe Les Républicains. pour le groupe Les Républicains. À partir du 22 janvier et pour une durée d’un mois, des centaines de pêcheurs français seront empêchés d’exercer leur activité dans le golfe de Gascogne – 600 navires sont concernés. Ce mois sans pêche, qui concerne les Français, mais non leurs collègues de l’Union européenne, a été proposé par le Gouvernement et durci par le Conseil d’État sous la pression des associations environnementales. Il s’agit de préserver les populations de petits cétacés des prises accidentelles. Ce mois sans pêche, c’est un nouveau coup porté à toute une filière qui, depuis des années, tente de surmonter un à un les obstacles qui se dressent devant elle. Entre les conséquences du Brexit, notamment la mise en place d’un plan de sortie de flotte, l’envolée des prix du gazole, des quotas de plus en plus restrictifs et des importations en hausse constante, c’est bien la pêche française qui qui est désormais en voie de disparition. Nos marins, leurs familles et, demain, toute la filière halieutique vont continuer de souffrir, malgré tous les efforts consentis depuis trente Ils s’équipent progressivement pour pallier toutes les contraintes qu’on leur impose. L’incompréhension les gagne : ne veut on pas valoriser le travail ? Ils sont empêchés de travailler Et, paradoxe naissant, en Bretagne, on réfléchit à importer par avion du poisson pêché à 8 000 kilomètres de nos côtes ! La plateforme d’indemnisation qui a été mise en place pour compenser le manque à gagner subi par les pêcheurs atténuera partiellement la douleur : elle ne concernera pas toute la filière ni ne guérira la maladie. Compenser n’est pas une perspective d’avenir. Monsieur le Premier ministre, après l’industrie et l’agriculture, voilà encore, avec la pêche, un fleuron français – garant de notre autonomie – qui souffre. Il est grand temps de changer de cap ! Qu’avez vous à dire aux pêcheurs et à leurs familles ?

La parole est à Mme Nadia Sollogoub, pour le groupe Union Centriste. Monsieur le président, mesdames, messieurs les ministres, mes chers collègues, ma question s’adresse à M. le ministre de l’agriculture Voilà un an exactement, un texte était adopté à l’unanimité des deux chambres. Ici, au Sénat, au cours de la discussion générale précédant son adoption, Olivier Dussopt, alors ministre du travail, avait dit, au nom du Gouvernement Nos agriculteurs et nos agricultrices, plus largement les Français et les Françaises, nous attendent sur cet horizon de justice sociale. » Ce texte, c’était la proposition de loi visant à calculer la retraite de base des non salariés agricoles en fonction des vingt cinq années d’assurance les plus avantageuses, et non plus sur l’ensemble de la carrière. question, promulguée le 13 février 2023, comporte un article unique, qui dispose que, dans un délai de trois mois à compter de sa promulgation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport précisant les modalités de sa mise en œuvre. prévu doit présenter notamment « le détail des scénarios envisagés et des paramètres retenus pour [son] application […] ainsi que, le cas échéant, les dispositions législatives et réglementaires qu’il convient de modifier ». Bref, ce rapport doit donner tous les éléments qui permettront à la Mutualité sociale agricole (MSA) de commencer cet énorme chantier. Or, à ce jour, un an après, aucun rapport ! Dès lors, les associations professionnelles agricoles et la MSA alertent sur le fait que, dans ces conditions, le dispositif ne sera probablement pas opérationnel dans le délai prévu par la loi. Monsieur le ministre, je relaie aujourd’hui cette alerte

du 23 juillet 2010 prises pour son application, la commission des lois a émis, lors de sa réunion de ce jour, un avis favorable, par 31 voix pour et 2 voix contre, à la nomination de Mme Marie Laure Denis à la présidence de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. L’ordre du jour appelle la désignation des vingt trois membres de la commission d’enquête portant sur la production, la consommation et le prix de l’électricité aux horizons 2035 et 2050. En application de l’article 8 alinéa 5, de notre règlement, les listes des candidats présentés par les groupes ont été publiées. Ces candidatures seront ratifiées si la présidence ne reçoit pas d’opposition dans le délai d’une heure prévu par notre règlement. groupe Les Républicains, l’examen de la proposition de résolution visant à condamner l’offensive militaire de l’Azerbaïdjan au Haut Karabagh et à prévenir toute autre tentative d’agression et de violation de l’intégrité territoriale de la République d’Arménie, appelant à des sanctions envers l’Azerbaïdjan et demandant la garantie du droit au retour des populations arméniennes au Haut Karabagh, présentée, en application de l’article 34 1 de la Constitution, par MM. Bruno Retailleau, Gilbert Luc Devinaz et plusieurs de leurs collègues

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, il y a plus d’un siècle, les mots suivants ont été prononcés tout près d’ici, à la Sorbonne : « C’était notre sœur d’Orient qui mourait, qui mourait parce qu’elle était notre sœur et pour le crime d’avoir partagé nos sentiments, d’avoir aimé ce que nous aimons, pensé ce que nous pensons, pensons, cru ce que nous croyons. » Ces phrases si justes, si émouvantes, ont été prononcées, quelques mois après le génocide arménien, par Anatole France. C’était en avril 1916.

affamée. En trois jours seulement, plus de 120 000 personnes – femmes, enfants, hommes et vieillards – ont été jetées sur les routes d’un exode peut être définitif.

effacés en trois jours seulement ! C’est la raison pour laquelle nous avons décidé de déposer cette résolution, que j’ai coécrite notamment avec

grave : la remise en cause de la souveraineté territoriale de l’Arménie. Notre objectif est de crier haut et fort notre opposition. Il est de dire que nous n’accepterons pas l’inacceptable, que nous n’admettrons pas l’inadmissible.

le voyage de Mme von der Leyen, qui est allée signer un accord gazier à Bakou. On sait parfaitement que cet accord gazier visait, en réalité, à contourner les sanctions pourtant décidées

constant de la Turquie, d’un espace commun néo ottoman, qui irait de la mer Égée à la mer Caspienne. D’où cette idée d’un couloir de Zanguezour, qui permettrait d’assurer une continuité territoriale pour cet espace.

nombreuses nations occidentales qui se sont déshonorées. Je me félicite que la France ait été l’une des rares nations à protester – peut être timidement, sans doute tardivement.

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, après l’offensive éclair des forces de l’Azerbaïdjan le 19 septembre dernier, pour la première fois depuis plus de deux mille ans, la quasi totalité des habitants de la république d’Artsakh a fui l’Arménie. Les seuls qui restent sont dans leurs tombes, d’ailleurs profanées dans des mises en scène absolument odieuses et lamentables, sans aucune protestation de la communauté internationale. Cet exode, vécu comme une nouvelle tragédie par tous les Arméniens, s’inscrit dans le conflit séculaire marqué par le génocide de 1915. Cette tragédie aurait pu être évitée. Le a récemment écrit, à propos de ce drame, que « presque personne ne l’avait vu venir ». Quelle hypocrisie ! Quelle contre vérité ! Les Arméniens, ainsi que ceux qui, comme nous, dans cet hémicycle ou dans celui de l’Assemblée nationale, ont suivi le conflit avaient prévenu depuis longtemps que cela arriverait. C’était même le projet que l’Azerbaïdjan et la Turquie avaient en tête. pas une année je n’ai cessé, à vos côtés ou aux côtés des députés et des sénateurs, d’alerter sur ce massacre annoncé. Nous connaissons tous la situation géopolitique de cette région, qui vit avec les attaques, les résolutions et des négociations qui s’enlisent depuis des dizaines d’années. Nous avons tous vu le conflit, que certains croyaient gelé, regagner de la vigueur en 2020. Nous avons tous été témoins de l’escalade, dans la solitude et l’indifférence pour les Arméniens. Aujourd’hui, nous voyons le drame qui se joue dans le Caucase. Nous avions d’ailleurs alerté, dans cet hémicycle, notamment à l’occasion de nos résolutions pour l’Arménie et l’Artsakh, en novembre 2020

de notre commission, Christian Cambon, du président du groupe d’amitié France Arménie, Gilbert Luc Devinaz, à qui je veux rendre hommage, des présidents de l’ensemble des groupes, au premier rang desquels, bien sûr, figure Bruno Retailleau, qui s’est investi personnellement, avec beaucoup d’énergie, de courage et de conviction. Le 7 juillet 1923 naissait la république autonome d’Artsakh, peuplée essentiellement d’Arméniens chrétiens, au sein de la République socialiste soviétique d’Azerbaïdjan, dont la population était principalement azérie, turcophone et chiite. Un siècle plus tard, le 28 septembre 2023, les dirigeants de l’Artsakh annonçaient la dissolution de l’entité indépendante de fait depuis 1991, avant d’être arrêtés par les forces azerbaïdjanaises. Pourtant, à l’été 2022, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, s’était rendue à Bakou afin de signer un accord honteux sur la livraison du gaz de l’Azerbaïdjan à l’Europe. Par la suite, elle a plusieurs fois loué ce pays comme un « partenaire énergétique fiable » de l’Union européenne. Quelle déroute morale, quelle honte et quelle infamie pour l’Europe et tous les pays qui l’ont soutenue ! Quelques mois plus tard, encouragé par ce soutien, l’Azerbaïdjan a lancé une attaque, non sur le Haut Karabagh, mais sur plusieurs zones à l’intérieur même de l’Arménie, du territoire souverain de ce pays reconnu par la communauté internationale, avec des frontières bien définies. Depuis lors, l’Azerbaïdjan occupe plus 100 kilomètres carrés de territoires incontestés et internationalement reconnus. En décembre 2022, il a imposé un blocus sur le couloir de Latchine, l’unique passage entre l’Artsakh et l’Arménie. En février 2023, la Cour internationale de justice de La Haye a émis une ordonnance contraignante, selon laquelle l’Azerbaïdjan devait immédiatement permettre la libre circulation des personnes et des marchandises dans le couloir l’Azerbaïdjan l’a ignorée, méprisée. Durant l’été 2023, la situation a empiré pour les 120 000 Arméniens du Haut Karabagh, avec de graves pénuries de nourriture, de combustibles et de médicaments. La malnutrition a sévi et la situation est devenue si critique que plusieurs organisations ont mis en garde contre un possible génocide par la faim et par le manque de soins. En août 2023, Luis Moreno Ocampo, ancien procureur de la Cour pénale internationale, a déclaré que les agissements de l’Azerbaïdjan devaient être considérés comme un génocide au regard de la convention sur ce crime. Pendant les plus de neuf mois qu’a duré le blocus, plusieurs dirigeants l’ont condamné et ont demandé à l’Azerbaïdjan d’y mettre J’ai encore en tête les images du président de notre groupe, Bruno Retailleau, sur place, aux côtés de plusieurs élus et de camions humanitaires bloqués par les forces azerbaïdjanaises, aux portes de l’Artsakh. Toutefois, contrairement à nos demandes, il n’y a eu ni sanctions ni même commencement de menace de sanctions. Là encore, quelle déroute morale ! Le gouvernement azéri a bien retenu le message : oui, il est possible de provoquer une crise humanitaire envers plus de 100 000 personnes, jusqu’à frôler le génocide, sans rien subir d’autre que des communiqués de presse timides des instances internationales ! Oui, il est possible de pratiquer la diplomatie du chantage. Oui, il est possible d’être un État corrupteur et corrompu. Tout est possible et tout se passe bien… Malheureusement, ce qui est valable pour l’Ukraine, à juste titre, ne l’a jamais été pour l’Arménie. Or, nous le savons tous, les mots n’ont jamais suffi à stopper les plans agressifs, génocidaires et barbares des États autoritaires. Des mesures beaucoup plus fermes étaient et seront nécessaires. L’Azerbaïdjan considère qu’elle n’a jamais forcé les populations à fuir, mais ces exodes expéditifs s’expliquent par la crainte justifiée de vivre sous le régime autocratique de M. Ilham Aliev, dont la famille règne à Bakou depuis 1993. Ce dictateur n’a jamais caché ses intentions génocidaires. Après le blocus du corridor de Latchine, après

Voilà désormais l’Arménie qui a la lourde tâche d’accueillir, de soigner et de rassurer seule 100 000 personnes ayant quitté leur pays, leur terre, leur foyer, dans une indifférence presque générale, après avoir vécu le pire. Je tiens à évoquer ici la mémoire des prisonniers torturés. Et je veux avoir une pensée pour Anouch Apetian, violée, démembrée, filmée, dont personne n’a parlé. Je n’ai entendu aucune association féministe parler du sort de cette femme ni d’autres, de l’indifférence… Dans ce contexte, alors qu’il cherchait à se rendre en Arménie, Ruben Vardanian, humanitaire arménien et ancien ministre d’État, a été illégalement arrêté. Il fait partie des derniers habitants d’Artsakh récemment arrêtés de manière arbitraire pour des raisons politiques et détenus illégalement. C’est également le

De nombreux autres Arméniens continuent d’être illégalement détenus dans les geôles de Bakou. Le peu d’informations accessibles sur leur état de santé et leur bien être est profondément inquiétant. On sait qu’ils subissent tortures et menaces. Ces personnes sont détenues en violation flagrante du droit international. Les conditions de leur détention sont particulièrement préoccupantes. Il faut conclure, ma chère

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, avec Bakou, « nous partageons les mêmes valeurs » et « l’énergie n’est que l’un des domaines dans lesquels nous pouvons renforcer notre coopération avec l’Azerbaïdjan et j’ai hâte d’exploiter tout le potentiel de notre relation Voilà des propos insupportables, que la France aurait dû dénoncer ! Monsieur le ministre, ils auraient pu être tenus par votre collègue ministre de la culture, Mme Dati, qui siège dans des associations affiliées à l’Azerbaïdjan, mais ce sont ceux de la présidente de votre Commission européenne, Mme Ursula von der Leyen. L’an dernier, par sa faute, le contribuable européen a versé près de 16 milliards d’euros à l’Azerbaïdjan, en vertu d’un contrat gazier signé en 2021 avec un autocrate qui, à l’époque, avait déjà le sang de 6 000 Arméniens sur les mains. Voilà dix jours, les montagnes d’Artsakh sont restées silencieuses. Les cloches des églises n’ont pas tinté dans la nuit de Noël, comme elles le faisaient pourtant depuis 1 700 ans. Une épuration ethnique, culturelle et religieuse a eu lieu 120 000 Arméniens d’Artsakh ont été déplacés, laissant derrière eux leurs maisons, leurs cimetières, leurs montagnes, leur terre. Ils ont été « chassés comme des chiens », comme l’avait promis Aliev. Depuis 2016, de graves heurts se succédaient déjà aux frontières de l’Artsakh et de l’Arménie, sans aucune réaction de notre part. En 2020, nous avons laissé passer la première agression armée massive de l’Azerbaïdjan. 2022, impuni et même promu au rang de partenaire, celui ci a bloqué le corridor de Latchine, sans que qui que ce soit ait eu la volonté de débloquer la situation. Personne n’a finalement été surpris de voir Aliev envahir l’Artsakh en 2023. Le 1 janvier de cette année 2024, la République d’Artsakh a cessé d’exister, et notre gouvernement, malgré un timide soutien de dernier instant à l’Arménie, semble avoir accepté cet Anschluss. en décembre 2022, Aliev, le complice et bras armé du sultan Erdogan, ne cachait pas son but, en affirmant : « Aujourd’hui, l’Arménie est notre territoire. La suite de l’engrenage mortel est l’ouverture du corridor du Zanguezour entre l’Azerbaïdjan et le Nakhitchevan, qui n’est rien d’autre que l’invasion du sud de l’Arménie. En découleront l’isolement de l’Arménie dans l’étau panturc et son affaiblissement, avant sa disparition finale. Plus nous attendons, plus nous la rendons inéluctable. C’est pourquoi la France doit boycotter la COP21 prévue à Bakou en décembre prochain et interrompre officiellement le processus d’adhésion de la Turquie à l’Union européenne. Les signaux diplomatiques doivent être clairs,

Les envahisseurs azerbaïdjanais ont bombardé la périphérie d’un village situé non loin de Goris. Un verger planté par les bénévoles de SOS Chrétiens d’Orient, auxquels je veux rendre hommage, a également été la cible de cette attaque. Ce bombardement a fait de nombreuses victimes parmi les civils arméniens.

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, en pleine période de vœux, on peut dire que 2024 commence sous de tragiques auspices. La guerre entre Israël et le Hamas se poursuit et pourrait conduire à un embrasement de la région. La guerre d’agression que la Russie de Poutine livre à l’Ukraine ne faiblit pas non plus. Malgré la résistance héroïque du peuple ukrainien, l’incertitude du soutien international fait redouter une victoire de la Russie. Celle ci serait un drame pour les Nations démocratiques. Les élections américaines risquent de fragiliser encore davantage la paix mondiale. Aucun pays ne dispose plus des moyens de préserver la paix. Ce morcellement des puissances semble raviver les conflits. Cette succession de guerres ne doit pas nous faire oublier celle qui a été menée par l’Azerbaïdjan contre l’Arménie pour le contrôle du Haut Karabagh. En 2020, une première agression de l’Azerbaïdjan, soutenue par la Turquie, s’est achevée par un accord de cessez le feu sous l’égide de Alors que la Russie s’est embourbée en Ukraine, l’Azerbaïdjan a repris l’offensive en 2023 pour prendre le contrôle total du Haut Karabagh, conduisant à l’exode des populations. Ces actions contreviennent gravement au droit international. Nous ne pouvons que les condamner. Malheureusement, l’Europe n’a pas encore su faire entendre sa voix ni assurer la paix. Alors que les conflits continuent de proliférer, nous devons lutter pour défendre nos valeurs et nos principes. Le droit des peuples à disposer d’eux mêmes, le multilatéralisme, la recherche de solutions négociées ne doivent pas devenir des vœux pieux. Ces valeurs sont au fondement d’un ordre international qui favorise la discussion plutôt que la coercition. Sans elles, il ne reste plus que le rapport de force. Bien sûr, l’Europe doit tenir compte de ses propres intérêts. La guerre en Ukraine et le soutien que nous apportons à Kiev mettent en exergue nos vulnérabilités, notamment énergétiques. Avec moins de gaz russe, nous avons besoin du gaz azerbaïdjanais, mais cela ne doit nous contraindre ni au silence ni à l’inaction. Aujourd’hui comme hier, nos compatriotes ont montré qu’ils étaient déterminés à contribuer à la souveraineté énergétique de notre pays et à renforcer notre indépendance. Collectivement, nous sommes parvenus à réduire notre consommation d’énergie primaire : voilà quatre ans que nous consommons moins qu’en 2019. C’est autant d’argent de moins pour les forces de l’obscurantisme Nous voulons nous donner les moyens de peser sur le cours de l’Histoire : nous devons bâtir maintenant notre autonomie stratégique. Nous ne devons pas reconnaître le résultat du coup de force de l’Azerbaïdjan. L’Arménie vit toujours sous la menace. Les regards se portent vers la Siounie, région qui fait figure de nouvelle cible. L’Azerbaïdjan pourrait tenter de s’y créer de force une continuité territoriale. Nous devons absolument éviter que de nouvelles atteintes ne soient portées à l’intégrité territoriale de l’Arménie. À cet égard, nous tenons à saluer l’action du Gouvernement, qui s’est notamment traduite par la livraison de matériel de défense.

Cette proposition vise aussi à appeler à mieux protéger l’Arménie contre les menaces qui pèsent sur elle. Elle tend enfin à permettre le retour des populations et la préservation du patrimoine culturel inestimable du Haut Karabagh. Plus que jamais, il est indispensable que l’Union européenne s’implique dans la résolution de ce conflit. L’Arménie ne doit pas être abandonnée. Nous le disons avec force et vigueur. Le groupe Les Indépendants soutiendra bien évidemment l’adoption de cette proposition

Manouchian symbolise à lui seul l’apport immense de la diaspora arménienne à notre pays. Peut être son entrée prochaine au Panthéon amènera t elle la majorité sénatoriale et le Gouvernement à jeter à l’avenir un regard moins caricatural et plus réaliste sur l’apport inestimable de l’immigration à notre pays Ainsi, nombre de membres de la communauté arménienne, à l’image de Manouchian, ont contribué très largement à faire rayonner la France, sa culture et ses valeurs. La singularité du lien qui nous unit à l’Arménie fait que l’injustice et l’horreur qui s’abattent sur les Arméniens du Haut Karabagh nous touchent particulièrement. Dans ce territoire, deux logiques s’affrontent : d’un côté, nous avons l’Azerbaïdjan, qui estime que tout soutien aux Arméniens du Haut Karabagh est une violation de son intégrité territoriale ; de l’autre, nous avons l’Arménie, qui appelle légitimement au respect du droit des peuples à l’autodétermination.

Depuis 2016 et la guerre des Quatre jours, Bakou n’a de cesse d’attaquer de façon périodique le peuple arménien du Haut Karabagh. L’offensive du 27 septembre 2020 a eu pour conséquence le massacre de 4 000 Arméniens en quarante quatre jours. Le 19 septembre dernier, une nouvelle offensive azérie a une nouvelle fois fait couler le sang dans le Caucase.

Malgré la tragédie qui s’abat sur ce territoire arménien ancestral, la communauté internationale peine à défendre les victimes du Haut Karabagh et à imposer une paix durable qui ne porterait pas préjudice au peuple arménien. d’une solution politique juste à ce conflit est rendue encore plus complexe par le jeu des différentes puissances régionales, lesquelles cherchent à étendre leur influence sur ce qu’elles considèrent comme leur pré carré. ajouter que la dépendance des pays européens aux énergies fossiles tend, par la force des choses, à aller de pair avec une dépendance politique vis à vis des pays qui nous fournissent ces énergies. En effet, la guerre en Ukraine a considérablement modifié la politique énergétique de l’Union européenne au bénéfice de l’Azerbaïdjan. En juillet 2022, la présidente de la Commission européenne s’est rendue à Bakou, afin de signer un protocole d’accord pour un partenariat stratégique dans le domaine de l’énergie. Les exportations de gaz vers l’Union européenne depuis Bakou ont augmenté de 40 % entre 2021 et 2022. Au regard de ce contexte et de notre dépendance énergétique, notre gouvernement sera t il libre demain de dénoncer les crimes commis contre le peuple arménien par l’Azerbaïdjan ? Je l’espère et le souhaite, monsieur le ministre. le ministre. Pour que la France retrouve sa voix singulière sur la scène internationale, il est important qu’elle garde comme boussole la défense des droits de l’homme. L’odeur du gaz ne doit pas nous aveugler au point d’oublier de dénoncer les atteintes à la dignité humaine et à la vie du peuple arménien. Enfin, mes chers collègues, ne tombons pas dans le piège de ceux qui voient ce conflit sous le prisme religieux et veulent nous entraîner dans une logique de guerre de civilisation ! Alors que les liens religieux, linguistiques, culturels et historiques de l’Iran avec l’Azerbaïdjan sont criants, l’Iran soutient pourtant l’Arménie.

l’hôtel de ville au centre du village. L’église ! Nous sommes dans un espace laïc, je n’utiliserai donc pas d’autre métaphore ! Monsieur le ministre, pour nous, écologistes, il n’y a pas de double standard et d’indignation sélective en fonction de nos émotions, de nos origines ou de nos affinités.

Nous dénoncerons toujours avec la même vigueur toutes les injustices, où qu’elles se produisent et d’où qu’elles viennent. Et nous déplorons de ne pas voir la même cohérence chez l’ensemble des responsables politiques. C’est pour toutes ces raisons que le groupe Écologiste – Solidarité et Territoires a cosigné et votera cette proposition de résolution, qui, je l’espère, redonnera dignité et respect au peuple arménien.

Madame la présidente, monsieur le ministre, madame l’ambassadrice, mes chers collègues, lorsque le Sultan voit que, pendant trois années, il a pu, grâce au sommeil complaisant de l’Europe, conduire impuni des massacres qui n’ont peut être pas de précédents dans les derniers siècles de l’histoire humaine, lorsqu’il voit l’Europe, se levant se levant dans le premier sursaut de ce réveil tardif, au lieu de se tourner vers les victimes du Sultan pour guérir leurs blessures, au lieu de se tourner vers les populations opprimées, pour les aider à conquérir leur indépendance, se faire d’abord, pour première démarche, pour première politique, la servante de ses intérêts à lui, il se dit qu’il tient l’Europe dans ses mains, qu’il peut, à son gré, jouer d’elle. Dès maintenant, vous l’avez investi de l’impunité de l’Europe. » Ainsi parlait Jean Jaurès le 15 mars 1897, depuis la tribune de la Chambre des députés, pour dénoncer l’indifférence coupable de l’Europe à la suite des massacres hamidiens. lustres plus tard, poursuivant l’œuvre exterminatrice du Sultan rouge, l’Azerbaïdjan a envahi le territoire de la République d’Artsakh et réduit toute sa population à l’exil. En trois jours, un État a disparu. En trois jours, des Arméniens ont tout quitté, pour ne laisser derrière eux que des infirmes et leurs morts. En trois jours, de nouveau dans l’indifférence générale, l’Azerbaïdjan s’est octroyé le droit de redessiner des frontières internationales et de procéder à un nettoyage ethnique qui a fait 120 000 victimes. De toute antiquité, le Haut Karabagh a été peuplé quasi exclusivement par des Arméniens. C’est un général britannique qui, le premier, en confia l’administration à un Azéri. Staline, par calcul, fragmenta davantage cette région, en rattachant à l’Azerbaïdjan les deux régions autonomes du Haut Karabagh et du Nakhitchevan. Néanmoins, la loi soviétique du 3 avril 1990 donnait la possibilité aux républiques et aux régions autonomes de faire sécession. C’est dans ce cadre juridique que la République d’Artsakh a proclamé son indépendance, qui a été ratifiée par référendum le 10 décembre 1991. chers collègues, les frontières de la République d’Artsakh sont des frontières internationales. En acceptant leur violation, nous avons consenti à la primauté de la force sur le droit et fragilisé l’intégrité territoriale de la République d’Arménie. Forte de son impunité, l’Azerbaïdjan exige maintenant une forme de souveraineté sur le Bas Karabagh, donc sur la province arménienne du Syunik, pour progressivement établir une continuité territoriale avec le Nakhitchevan et la Turquie. Si l’Union européenne et les instances internationales laissent impunie l’agression contre la République d’Artsakh, le Syunik sera annexé par l’Azerbaïdjan comme l’a été le Haut Karabagh. Pour protéger l’Arménie, il faut sanctionner l’Azerbaïdjan. Monsieur le ministre, il est du devoir de la France de tout mettre en œuvre auprès de ses alliés, des pays membres de l’Union européenne et de la Commission européenne pour qu’ils condamnent l’absorption de l’Artsakh et obligent l’Azerbaïdjan au respect intangible des frontières de l’Arménie. Par ailleurs, il est inacceptable qu’Israël, l’Italie, la Bulgarie, l’Espagne, la République tchèque, la Slovaquie et même l’Ukraine continuent de fournir à l’Azerbaïdjan des armes que ce pays retourne contre le peuple arménien. Ne vendons pas notre honneur contre un plat de lentilles en achetant le gaz et le pétrole azéris en échange de notre silence sur l’asservissement du peuple arménien Le Parlement européen, par sa résolution du 5 octobre 2023, a demandé à une très large majorité la suspension du protocole d’accord sur un partenariat stratégique dans le domaine de l’énergie. La France doit maintenant tout mettre en œuvre pour que cette suspension soit effective et pour que les avoirs des dirigeants azéris soient saisis, comme le prévoit la présente proposition en entrant dans cet hémicycle, vous pouvez passer devant le buste d’Auguste Scheurer Kestner, qui a été sénateur de 1875 à 1899. Pendant près de vingt cinq ans, il a été au sein de notre assemblée le représentant d’une Alsace annexée par l’empire allemand. Jusqu’à sa mort, il a entretenu l’espoir du retour, comme ces nombreux Alsaciens et Lorrains qui préférèrent l’exode pour garder leur nationalité française. Cette résolution doit être pour tous les Artsakhiotes un message de fraternité et d’espoir. Rien n’est jamais définitif, et les exils peuvent être provisoires. Sachez que nous demeurerons à vos côtés pour préserver votre droit, celui qu’a un peuple de disposer de lui même et de refuser l’asservissement

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, comme l’a dit le président Retailleau, nous sommes réunis pour condamner l’offensive militaire de l’Azerbaïdjan au Haut Karabagh et prévenir toute autre tentative d’agression et de violation de l’intégrité territoriale de la République d’Arménie sans doute avec retard, hélas ! L’inquiétude que nous partagions dans cet hémicycle le 25 novembre 2020 lors du débat sur la nécessité de reconnaître la République du Haut Karabagh a été confirmée par une offensive sanglante de l’Azerbaïdjan. Pour cette séance publique qui nous rassemble, j’aurais pu me contenter de reprendre le discours que j’avais alors prononcé. Je n’y ôterais aucun mot, aucune remarque, rien ! Je parlais d’urgence à agir, de devoir moral et d’exigence. Ces mots d’ordre gardent leur force plus que jamais, alors que le contexte international a changé et que l’Arménie se retrouve isolée, sous surveillance de la Russie et de la Turquie. Je rappelais la fierté qui était la nôtre quand la France avait su reconnaître le génocide arménien du 24 avril 1915. Que reste t il, mes chers collègues, de cette fierté ?

La République d’Arménie et le Haut Karabagh ont été victimes du cynisme de leurs voisins et – pardonnez moi par avance de la dureté de l’expression – de la lâcheté collective. Je l’affirme, le Haut Karabagh et ses habitants ont été sacrifiés dans un silence assourdissant de la communauté internationale. Oui, ils ont été sacrifiés sur l’autel d’intérêts économiques et géopolitiques. En premier lieu, évidemment, ceux qui sont liés à la crise de l’énergie et au jeu subtil de l’Azerbaïdjan, qui a su faire miroiter les avantages de ses réserves de gaz, alors que l’Europe tentait d’afficher sa condamnation de l’évasion de l’Ukraine par Moscou. Devrai je aussi regretter le jeu trouble d’Ankara, d’Erdogan, ravi d’affaiblir toujours plus Erevan ? Aussi, j’avoue ma honte, notre honte collective, la honte de la communauté internationale et – il faut le dire aussi – celle de l’ONU. Honte Honte à l’ONU, laquelle, chaque jour qui passe, ressemble toujours plus à sa grande sœur, la fameuse Société des Nations,

fait, vous me concéderez, monsieur le ministre, que désormais la confiance et le droit international ne semblent pas peser d’un grand poids face à la volonté expansionniste de dirigeants qui oscillent entre agressivité, bellicisme et populismes en tous genres. Rassurez vous, je ne m’engagerai nullement dans la lecture d’une liste exhaustive de ces personnalités. Je laisse aux juristes et aux diplomates aguerris le soin et la responsabilité de l’établir. Toutefois, devrions nous

Évitons leur ce triste travail, en portant avec fermeté et volonté notre message pour l’intégrité de l’Arménie. Car, mes chers collègues, si nous sommes comptables de ce fiasco aux lourds tributs humanitaires, pour les soldats, d’abord, et pour la jeunesse arménienne, ensuite, qui ont payé de leur sang les les assauts de l’Azerbaïdjan, sachons aussi faire entendre notre voix. Loin d’être purement symbolique, cette résolution permet de réaffirmer le soutien de la France à ce pays qui fait battre le cœur de la démocratie aux marges du Caucase. Dans un monde qui se fracture, où les haines attisent les conflits, notre voix doit se faire entendre pour accompagner, aider et soutenir un peuple qui marche sur le chemin du progrès – le peuple arménien, dont on connaît les souffrances, mais dont on sait aussi la richesse. Parce que nous respectons ce pays, parce que nous l’aimons et parce ce qu’il nous a apporté et continuera à nous offrir, soyons à ses côtés, sans états d’âme. C’est pour cela que le groupe RDSE, à l’unanimité, votera cette résolution. La

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous sommes réunis aujourd’hui pour évoquer un conflit international douloureux, aux répercussions dévastatrices, dont les racines s’enfoncent dans un passé lourd et complexe. La première guerre du Haut Karabagh, achevée en 1994 après plus de six années de conflit, a été suivie par une seconde guerre en 2020, qui a duré un mois. En décembre 2022, les forces armées azerbaïdjanaises ont créé un blocus total dans la région du Haut Karabagh. Elles ont pris le contrôle du corridor de Latchine et ont progressivement pris en étau la population du Haut Karabagh, privée d’importation de produits alimentaires et de médicaments, puis faisant face à une pénurie d’essence. Le 19 septembre 2023, l’Azerbaïdjan a violé le cessez le feu, conclu avec l’Arménie en 2020, en lançant une offensive militaire qui a pris fin le lendemain, le 20 septembre. La rapidité de ce conflit éclair ne doit pas minimiser l’ampleur de ses conséquences désastreuses, notamment géopolitiques. N’oublions pas que l’Arménie et l’Azerbaïdjan sont géographiquement très proches de la Russie et de l’Iran, deux États qui occupent déjà des rôles de premier plan dans d’autres conflits mondiaux. Très courte, cette guerre d’un jour a poussé l’Arménie à ratifier son adhésion à la Cour pénale internationale, une décision prise pour un affront par Moscou. Même si les combats sur le terrain ont cessé, nous devons rester vigilants. L’attaque azerbaïdjanaise a ravivé de vieilles tensions dans le Caucase, une région peuplée d’anciennes entités soviétiques. Par son offensive militaire, l’Azerbaïdjan a bafoué le droit à l’autodétermination du peuple arménien, principe garantissant son intégrité et sa sécurité. Par son agression, il a également révélé des intentions génocidaires et une volonté d’épuration ethnique. Outre ses velléités de conquêtes territoriales, il s’en il s’en est pris au riche patrimoine culturel et religieux arménien, comme pour effacer toute trace de l’existence du peuple arménien dans la région du Haut Karabagh. La présente proposition de résolution rappelle que toutes ces atteintes au peuple arménien constituent un crime contre l’humanité au regard du droit international. Ces atteintes à l’intégrité du peuple arménien sont intolérables. Nous condamnons unanimement l’offensive militaire menée par l’Azerbaïdjan dans la région du Haut Karabagh. Nous demandons tous que le droit international et l’intégrité du peuple arménien soient respectés. C’est en vertu de ces principes et au regard de la tragédie qui s’est déroulée au Haut Karabagh que cette proposition de résolution transcende les clivages partisans. Dans un contexte où l’attention internationale est captivée par des crises majeures au Proche Orient, en mer Rouge ou encore en Ukraine, il est impératif de rappeler le déroulé des événements tragiques du Haut Karabagh et de mettre en lumière le soutien continu de la France à la population arménienne touchée par ce conflit. En toute situation, la France s’engage aux côtés des populations injustement affectées par les conflits armés. En raison de l’opération militaire azerbaïdjanaise, près des deux tiers des 120 000 habitants du Haut Karabagh ont été contraints de fuir. Parmi eux, 30 000 enfants ont subi la guerre. Ces personnes sont devenues, du jour au lendemain, des réfugiés dans une situation de grande détresse. La majorité d’entre elles trouve refuge en Arménie, laquelle est débordée par cet afflux massif et dépassée par la tragédie humanitaire qui l’accable. La France va continuer de la soutenir, notamment grâce à l’aide d’urgence de 15 millions d’euros votée par le Parlement le 30 novembre 2023. Ce nouvel effort porte la contribution française à 27,5 millions d’euros pour l’année 2023. Il s’accompagne d’actions de solidarité de la part de la société civile et des collectivités territoriales françaises en faveur de la population arménienne et des réfugiés des réfugiés pris au piège dans l’enclave du Haut Karabagh, où ils ont enduré des souffrances inimaginables. Les populations déplacées doivent pouvoir retourner chez elles en toute sécurité. perspective, il est essentiel de respecter strictement l’intégrité territoriale et la souveraineté de l’Arménie, comme le dispose clairement la proposition de résolution. Nous exigeons également la libération inconditionnelle des prisonniers de guerre.

Ce texte vise à réclamer une réponse robuste de la France, de l’Union européenne et de la communauté internationale. Il nous invite collectivement à défendre les principes du droit international, du droit humanitaire et du droit à l’autodétermination des peuples. Ces droits et toutes les valeurs qu’ils expriment sont des fondements essentiels de nos démocraties, qui contribuent à la stabilité de l’Union européenne et de son voisinage. Leur respect est la seule voie possible vers une paix durable entre l’Azerbaïdjan et l’Arménie.

pourrait paraître décalé au vu des négociations qui ont été récemment entamées. Pourtant, cette avancée diplomatique ne doit pas cacher les tensions qui restent prégnantes dans la région. Le risque d’invasion du sud de l’Arménie ne s’est pas évaporé, et le sort réservé aux intérêts arméniens reste préoccupant. La préservation de la souveraineté nationale de ce petit pays du Caucase doit rester notre priorité. Le traumatisme de la Seconde Guerre mondiale a conduit à la mise en place collective d’instances

Mes chers collègues, je nous exhorte à ne pas nous y habituer ! Je nous souhaite de toujours porter haut l’étendard de la paix face à une sorte de fatalisme belliqueux. L’élimination ethnique est, rappelons le, la forme extrême de violence entre humains. Celle qui a eu lieu en Arménie ne peut être tolérée.

nommer les choses et mettre en exergue un conflit qui est depuis trop longtemps invisible, qui s’est transformé dans le Haut Karabagh en épuration ethnique territoriale.

Cette image est cependant sujette à caution, dans la mesure où elle nous donnerait trop facilement bonne conscience. En effet, lorsqu’elles ne sont pas sous le feu des médias et que la communauté internationale ne s’élève pas contre elles, les puissances belligérantes, portant souvent une vision impérialiste, peuvent avoir le sentiment que leurs actions se feront en toute impunité.

La montée des nationalismes est inquiétante. Elle favorise les revendications territoriales et l’extrémisme, qui est le vecteur naturel de la conflictualisation des relations. Les tendances nationalistes sont en train de submerger notre pays, ces idées mortifères n’étant plus réservées à l’extrême droite.

en ce domaine. Notre conception du droit international doit primer les nouveaux rapports de force qui nous sont imposés dans une logique d’impunité.

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, au carrefour des civilisations, le Caucase, « montagne des langues », est riche de sa diversité culturelle, religieuse, linguistique et ethnique. La région a connu au fil des siècles une histoire mouvementée, qui n’est pas sans lien avec les événements récents que nous condamnons. La période soviétique a garanti une certaine stabilité, mais au prix d’un verrouillage sécuritaire strict. Je rappelle qu’Heydar Aliev, premier président de l’Azerbaïdjan indépendant, avait été général du KGB ère a néanmoins complexifié la situation locale et n’a pas pu empêcher les premières tensions entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan, lesquelles ont ensuite dégénéré en conflit gelé, ponctué d’escarmouches et d’affrontements ouverts.

cette situation, puis l’Ukraine. Après 2008, l’Azerbaïdjan, qui s’était rapidement rapproché des Occidentaux et enrichi par le pétrole et par le gaz de la Caspienne, a bien reçu le message russe en revenant à de meilleurs sentiments à l’égard de Moscou. À qui voulait l’entendre, les Azerbaïdjanais n’ont jamais fait mystère de leur volonté de mettre à profit cette richesse pour améliorer le sort de leurs déplacés et pour récupérer, au besoin militairement, les territoires considérés comme perdus en 1994. Ce pari de long terme a été gagnant face à l’Arménie : privée de ressources naturelles et lâchée par les Russes, celle ci s’enfonçait dans la crise économique, exclue de fait du boom énergétique de la Caspienne. Le retour en force des ex empires comme la Turquie, liée culturellement à Bakou, et la Russie, en quelque sorte désinhibés dans l’usage de la force et dans la violation du droit, a facilité les récentes actions militaires azerbaïdjanaises. Cette guerre instrumentalisée devient une nouvelle zone de friction entre les Occidentaux que nous sommes et les partisans d’un nouvel ordre mondial fondé sur la dictature.

faire cesser la destruction méthodique du patrimoine historique. Tel est l’objet du texte de la résolution débattue aujourd’hui.

déplacement à Erevan, j’ai pu assister à la présentation aux membres de l’assemblée parlementaire de l’OSCE du plan de paix du Premier ministre arménien.

choisi la France pour leur première visite officielle à l’étranger. L’Azerbaïdjan est membre du Partenariat oriental de l’Union européenne, dont les parties se sont notamment engagées à défendre les valeurs fondamentales qu’elles partagent : renforcement de la démocratie et de l’État de droit, protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales… Comme la Russie, ce pays est un État participant à l’OSCE, organisation dont la raison d’être est la diplomatie préventive, la résolution pacifique

Les exportations des produits énergétiques azerbaïdjanais vers l’Union européenne devraient se maintenir, voire croître. Certains énergéticiens européens ont des intérêts directs dans la Caspienne ; leurs concurrents russes ou chinois ne seraient pas fâchés de les remplacer.

chers collègues, la diplomatie parlementaire est précieuse. Elle permet à des élus d’échanger en toute bienveillance, ainsi que de partager leurs espoirs, leurs doutes

J’exprime enfin ma reconnaissance aux présidents de l’ensemble des groupes politiques du Sénat. Ils ont accepté de cosigner ce texte, faisant la démonstration, par cette belle unanimité, que la cause arménienne dépasse les clivages politiques.

la défense de l’ordre international et de la diplomatie contre l’emploi de la force et le retour des logiques de puissance. Comme je l’indiquais il y a un instant, la diplomatie parlementaire a parfois une longueur d’avance sur la diplomatie officielle, grâce aux liens de confiance confiance et de fraternité qui se tissent entre parlementaires. Grâce à ces liens, nos amis députés arméniens nous ont livré avec une grande franchise leurs réflexions sur la situation de leur pays. À plusieurs reprises, notamment en 2019, ils nous ont alertés sur les risques d’une agression militaire. Leurs craintes étaient fondées. Nous les avons relayées auprès des autorités françaises, mais elles n’ont pas toujours été entendues, en tout cas pas assez tôt.

fait suite à l’offensive militaire menée par l’Azerbaïdjan en septembre dernier, en violation de l’accord de cessez le feu. En apparence, le contexte a évolué ces dernières semaines, avec la libération de trente deux prisonniers et la volonté affichée des deux pays de trouver une voie de conciliation. Nous soutiendrons bien sûr toute initiative allant dans le sens d’une paix équitable et sincère. Il n’en demeure pas moins absolument nécessaire de dénoncer ce qu’ont vécu et que vivent encore les 120 000 Arméniens d’Artsakh. Après plus de dix mois d’un blocus qui les a privés de tout, tous ont été contraints de quitter leur terre et leur maison. Ce que notre ancienne ministre des affaires étrangères a qualifié d’« épuration ethnique » a, en réalité, toutes les caractéristiques d’un véritable projet génocidaire. Comme l’exode contraint des populations n’était pas suffisant, le président Aliev est venu piétiner leur drapeau et effacer toute trace de leur présence Stepanakert, en détruisant le patrimoine arménien et en rebaptisant les rues du nom des auteurs du génocide de 1915. Ces actes odieux nous ont glacé le sang.

Nous ne pouvons nous y résoudre. Tel est le sens de la résolution qui vous est présentée, mes chers collègues. Premièrement, elle vise à condamner l’offensive militaire de septembre dernier, condamnation dont il devrait logiquement résulter l’application d’un régime de sanctions au niveau européen européen et international. Deuxièmement, elle tend à appeler à la libération immédiate des autorités politiques démocratiquement élues du Haut Karabagh ainsi que de tous les prisonniers de guerre. Troisièmement, elle a pour objet de souligner l’impérieuse nécessité de garantir aux populations arméniennes du Haut Karabagh un droit au retour en toute sécurité. Quatrièmement, la résolution vise à alerter sur les menaces qui pèsent sur le patrimoine arménien du Haut Karabagh. Cinquièmement, et enfin, l’Arménie doit avoir les moyens de se défendre pour prévenir toute nouvelle tentative d’agression

ne rien lâcher et résister, malgré les menaces, les peurs et le désespoir. Alors que Missak Manouchian entrera dans quelques semaines au Panthéon pour avoir défendu les valeurs de notre pays et de notre république, nous nous devons à notre tour de défendre la République d’Arménie et les valeurs démocratiques qu’elle incarne dans cette région tourmentée du Caucase, voisine de l’Europe.

L’Arménie doit pouvoir protéger sa population et son territoire, et notre pays continuera à agir dans ce domaine dans un esprit de responsabilité et sans aucun esprit d’escalade. Dans la même logique politique, nous renforcerons notre présence dans la région par l’ouverture prochaine d’une agence consulaire et nous continuerons à appuyer le développement de projets d’infrastructures dans les domaines stratégiques, tels que les transports, l’énergie et l’eau.

À la demande de la France, le Conseil des affaires étrangères a décidé d’accroître les effectifs de la mission civile de l’Union européenne en Arménie. Il s’agit de renforcer pour nous la présence européenne sur les points sensibles de la frontière entre ce pays et l’Azerbaïdjan.

Ces avancées sont essentielles. Nous nous en félicitons. Vous pouvez compter sur notre détermination pour continuer à faire bouger les lignes. Mesdames, messieurs les sénateurs, la conviction de la France reste inchangée : seul un processus négocié apportera la paix aux populations du Sud Caucase. La France souhaite que les négociations se poursuivent pour normaliser les relations entre les deux États. Elle apporte tout son soutien aux discussions et aux efforts de médiation, à la fois européens et américains. Il est important que l’Azerbaïdjan lève toute ambiguïté sur le respect de l’intégrité territoriale de l’Arménie. Nous souhaitons que le Caucase et le Sud Caucase soient un espace de paix et de coopération, où les frontières sont ouvertes. Ce serait un signal très fort, y compris pour nos relations avec les pays de la région.

positif, mais insuffisant. Espérons que de telles annonces constituent un premier pas pour résoudre la situation des autres détenus, que vous avez tous évoquée. Ma conviction est aussi qu’une paix juste et durable se trouve possible uniquement dans le respect du droit international, de la souveraineté, de l’intégrité territoriale et de l’inviolabilité des frontières des deux États. Nous serons intransigeants sur ces grands principes. outre, l’Azerbaïdjan doit prendre toutes les mesures nécessaires pour empêcher et pour punir les actes de dégradation et de profanation du patrimoine culturel, religieux et funéraire arménien.

Mesdames, messieurs les sénateurs, telle est la ligne de conduite de la France. Avec constance et exigence, nous œuvrerons pour la paix, soutiendrons tous les efforts sincères en faveur de cette dernière, défendrons le droit international

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues,

L’actualité nous rappelle brutalement, souvent, hélas ! à la suite du tragique suicide d’un jeune, la souffrance psychique de nombreux enfants, adolescents et étudiants.

Oui, de plus en plus de jeunes connaissent un état dépressif. Si les causes du mal être sont propres à chaque individu et parfois complexes à établir, les études sur la santé mentale recensent plusieurs marqueurs.

L’isolement concerne plus particulièrement les étudiants, qui sont souvent coupés de leurs proches. C’est très anxiogène, en particulier en milieu urbain. Nous l’avons mesuré durant la pandémie de la covid Les violences morales, physiques ou sexuelles au sein de la famille, ou en dehors de celle ci, sont également à l’origine de drames et de nombreux troubles psychiques. Concernant les violences extrafamiliales, la question du harcèlement scolaire tourmente des milliers d’enfants et hante des parents souvent impuissants face à ce phénomène, quand ils ne sont pas tout simplement ignorants de la tragédie qui s’immisce sournoisement dans leur foyer. La semaine dernière encore, un jeune Toulousain, victime de harcèlement scolaire, s’est poignardé en plein cours. On le constate et on le déplore, le harcèlement scolaire a pris une tournure encore plus dramatique depuis son irruption sur les réseaux sociaux. Longtemps cantonné aux cours d’école, il trouve une audience démultipliée et extrascolaire sur les réseaux, qui ne fait qu’aggraver le phénomène pour les victimes.

Quant au changement climatique, il provoque aujourd’hui ce que l’on appelle l’éco anxiété, un mélange de peur, de colère et de tristesse pouvant déboucher aussi sur des états dépressifs. À ce sombre tableau, il faut ajouter les inégalités qui affectent les jeunes différemment selon leur milieu social ou même leur genre. À l’évidence, la précarité est un facteur de dégradation de la santé mentale, les difficultés financières constituant une préoccupation qui peut tourner à l’anxiété et, en parallèle, constituer un handicap pour l’accès aux soins. En Nouvelle Aquitaine, par exemple, un jeune sur quatre n’a pas de médecin traitant. Concernant les inégalités de genre, les études sur les troubles psychiques soulignent que, en raison de la prévalence des violences faites aux femmes, la dépression touche davantage les jeunes filles. Tous ces facteurs aboutissent à un constat clinique dramatique : troubles du sommeil, phobie scolaire, anorexie, troubles obsessionnels compulsifs, dépression, schizophrénie, consommation abusive d’alcool, drogue, agressivité et actes suicidaires dans les cas les plus tragiques. Mes chers collègues, les chiffres fournis par Santé publique France sont glaçants. En 2021, près de 43 % des étudiants ont déclaré s’être retrouvés en situation de détresse psychologique, contre 29 % l’année précédant la pandémie de covid Alors que la dépression touchait déjà 11,7 % des 18 24 ans en 2017, en 2021, ce sont 21 % des jeunes, soit le double, qui sont tristement concernés. En septembre 2023, soit près de deux ans après les difficiles périodes de confinement, les passages aux urgences pour gestes et idées suicidaires, troubles de l’humeur et anxiété ont nettement augmenté chez les enfants de moins de 18 ans, avec un corollaire inquiétant, l’augmentation de la consommation médicamenteuse : près de 5 % d’enfants ingèrent des psychotropes. Depuis 2014, la prescription d’antipsychotiques, d’hypnotiques, de sédatifs et d’antidépresseurs ne cesse d’augmenter. Face à cette situation, quelles réponses apporter ? Au regard de son ampleur, ce fléau nécessite une prise de conscience collective et une action publique volontaire et ambitieuse. Tel est d’ailleurs le sens d’une déclaration en juin 2022 de la Défenseure des droits, qui invitait le Gouvernement à mettre en place un plan d’urgence pour la santé mentale des jeunes face à la gravité de la situation. Dans cet hémicycle, en réponse à la question d’actualité que j’évoquais au début de mon propos, le ministre de la santé et de la prévention d’alors rappelait que « la santé mentale, particulièrement celle des jeunes, doit être une priorité pour ce gouvernement

lorsqu’on leur annonce qu’il leur faudra attendre deux ans pour obtenir une place dans un centre médico psycho pédagogique (CMPP). Pourquoi ces délais ? Parce que nous comptons seulement 600 pédopsychiatres pour près de 10 millions d’enfants et 800 médecins scolaires, soit un médecin pour 15 000 élèves. En outre, l’offre d’équipements ambulatoires et hospitaliers du secteur infantojuvénile est répartie de façon inégalitaire sur le territoire. Ces établissements sont dépassés par les demandes, d’autant plus que les familles n’y avancent pas les frais. les frais. Au manque de professionnels de santé spécialisés et de places en milieu médical s’ajoute le problème de l’inadaptation des soins pour les jeunes patients, faute de moyens pour une approche globale. Ce défaut de prise en charge peut conduire à des situations de surmédication pour des milliers d’enfants, qui sont traités avec des produits normalement destinés aux adultes. Sans vouloir diaboliser le recours aux médicaments, qui, dans nombre de cas, est nécessaire pour soutenir les jeunes patients, il apparaît indispensable qu’un effort soit entrepris pour renforcer le déploiement des pratiques psychothérapeutiques et de prévention, afin de constituer une offre robuste de soins de première ligne et d’éviter la médication. Je ne dis pas bien sûr, madame la ministre, que rien n’a été réalisé, et les quelques dispositifs qui ont fait leurs preuves au cours de ces dernières années doivent être poursuivis et renforcés. Je pense à MonParcoursPsy pour les moins de 18 ans, aux maisons des adolescents, aux points santé dans les missions locales, au Fil Santé Jeunes d’aide à distance, aux campagnes nationales de sensibilisation, telles que « En parler, c’est déjà se soigner », ou au dispositif de recontact VigilanS, qui vise à prévenir les tentatives de suicide.

Parce que les troubles mentaux apparaissent très tôt dans la vie – la moitié des pathologies s’installe avant l’âge de 18 ans –, j’attire également votre attention, madame la ministre, sur le rôle de la médecine scolaire.

Je n’ignore rien des problèmes de démographie médicale, mais il est urgent de repenser les missions et de renforcer les moyens du service de santé scolaire pour le rendre plus performant et plus attractif pour les médecins et les infirmiers.

promouvoir dans les discours la nécessité d’une France résiliente est vaine si, dans le même temps, on ne donne pas à chaque enfant le moyen de forger sa propre résilience et de faire respecter ses droits élémentaires. de cette proposition de résolution, nous invitons le Gouvernement à ériger la santé mentale des jeunes en grande cause nationale, à donner de la visibilité à ce fléau et à briser ce tabou. Nos jeunes en difficulté ont besoin d’une prise en charge précoce et de qualité, de meilleures capacités d’accueil en soins de psychiatrie et d’accès aux psychologues, d’une médecine scolaire à la hauteur des besoins et d’une prise en charge psychothérapeutique autant que cela

de saluer, dans notre tribune d’honneur, une délégation conduite par Mme Annita Demetriou, présidente de la Chambre des représentants de Chypre. Elle est accompagnée par notre collègue Pascale Gruny, en remplacement de Samantha Cazebonne, présidente du groupe interparlementaire d’amitié France Chypre. La délégation a été entendue ce matin par la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, puis elle a été reçue en audience par le président du Sénat, Gérard Larcher. La France entretient d’excellentes relations bilatérales avec Chypre, fruit de notre histoire, mais aussi au sein de l’Union européenne, que ce pays a rejointe en 2004. Nous nous réjouissons de la perspective du renforcement de nos coopérations en matière de défense et en Méditerranée orientale. Mes chers collègues, en votre nom à tous, permettez moi de souhaiter à Mme Annita Demetriou et à la délégation chypriote la plus cordiale bienvenue au Sénat, ainsi qu’un excellent et fructueux séjour ! Nous reprenons

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, le suicide est l’une des premières causes de mortalité chez les 15 24 ans. Entre 2020 et 2021, une explosion des syndromes dépressifs a été observée chez les jeunes, ainsi qu’une augmentation du nombre des tentatives de suicide, notamment chez les moins de 15 ans. Nous ne pouvons pas accepter que des personnes à l’aube de leur vie en arrivent à perdre, à ce point, toute confiance en l’avenir. Bien sûr, la crise sanitaire a eu un effet désastreux sur l’équilibre psychologique des jeunes et ses conséquences sont encore bien réelles aujourd’hui, les addictions liées au manque de perspectives, au stress ou au désespoir Cependant, il serait imprudent de justifier les difficultés de la jeunesse par la seule persistance des effets des confinements successifs et de la désocialisation qui en a résulté. Les causes de la dégradation de leur état de santé psychique sont multiples et complexes et s’enchevêtrent parfois. Le passage à l’adolescence peut être une période particulièrement difficile et cette longue transition vers l’âge adulte peut sembler insurmontable pour certains jeunes. Les violences intrafamiliales, qui ont explosé durant la crise sanitaire, ont aussi eu un rôle prépondérant dans l’évolution de la santé psychique des jeunes. Que l’enfant en soit victime directement ou indirectement, elles représentent un traumatisme qui aura de très lourdes répercussions sur sa vie et sur son équilibre.

Le nombre croissant et alarmant d’étudiants ayant recours à l’aide alimentaire ne peut nous laisser indifférents. La précarité, qui mène souvent à l’isolement, est un facteur indéniable de troubles psychologiques. Je rappellerai également les effets des réseaux sociaux, dont la nocivité n’est plus à démontrer depuis l’avènement des smartphones, qui permettent aux jeunes d’être connectés en permanence, bien souvent avec des amis virtuels. Toutes les études sur le sujet en attestent : plus un jeune passe de temps sur certaines applications, plus les conséquences délétères sur sa santé mentale sont importantes. Il faut enfin citer le harcèlement scolaire, lourdement aggravé par les réseaux sociaux, dont 800 000 à 1 million d’enfants sont victimes chaque année. Notre groupe est d’ailleurs très investi sur ce sujet, sur lequel notre ancienne collègue Colette Mélot avait publié un excellent rapport d’information en 2021. J’espère que la ministre de l’éducation nationale nouvellement nommée saura poursuivre ce combat prioritaire, afin que nous n’ayons plus à déplorer de suicides liés au harcèlement scolaire, de tels drames étant épouvantables. L’école a un rôle majeur à jouer dans la détection des altérations de la santé mentale chez les jeunes. Plus les troubles sont détectés tôt, plus les chances de guérison augmentent. Cependant, la médecine scolaire est en très grande difficulté. Le nombre de médecins scolaires a baissé de 20 % en dix ans, et seuls 20 % des élèves ont eu accès à la visite médicale obligatoire de la sixième année, selon un récent rapport d’information de l’Assemblée nationale. La détection des troubles de santé mentale n’est pas à la hauteur des enjeux, et le risque est qu’un certain nombre d’enfants et d’adolescents ayant échappé aux actions de prévention ne se retrouvent dans un parcours de soins psychiatriques quelques années plus tard. Le Gouvernement nous explique que les moyens ne manquent pas : les postes existent, mais ils ne sont pas pourvus, le taux de couverture étant d’à peine 50 %. Ce problème d’attractivité dissimule une question de revalorisation de la fonction, même s’il faut admettre que le manque de médecins concerne effectivement la majeure partie du territoire, et non pas seulement le secteur

L’Essonne n’est pas épargnée par la désertification médicale. Le manque de personnels dans le secteur psychiatrique est criant, comme me l’a confirmé le chef du pôle psychiatrie de groupe hospitalier Nord Essonne. Allouer des moyens supplémentaires à la prise en charge au long cours des jeunes est indispensable. Cela passe par le recrutement de médecins, y compris étrangers, d’infirmiers formés en psychiatrie et de psychologues. Cela suppose également de favoriser l’internat dans la discipline et de rendre le métier plus attractif. En un mot, il s’agit de redonner du sens La prise en charge en psychiatrie infante juvénile est également l’une des missions de l’établissement public de santé Barthélemy Durand dans l’Essonne. Celui ci offre un ensemble de structures de soins réparties territorialement permettant d’articuler actions de prévention et actes de soins au plus près de l’environnement familial et social des personnes.

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, je veux, au nom du groupe Union Centriste et de mon collègue Olivier Henno, que je remplace aujourd’hui, saisir l’occasion de cette proposition de résolution pour formuler quelques observations et remarques sur l’accès aux soins dans notre pays et, plus largement, sur la prise en charge en psychiatrie. de Nathalie Delattre d’ériger la santé mentale des jeunes en grande cause nationale. C’est un fait avéré et indiscutable que les jeunes Français sont de plus en plus anxieux. Les causes sont multiples. impossible de ne pas évoquer la crise du covid 19 et le confinement. Des jeunes isolés, enfermés et privés de relations sociales peuvent légitimement revendiquer une souffrance psychologique

il ne s’agit pas là des seules causes de l’anxiété dont souffre une partie de la jeunesse française. Les guerres en Ukraine et en Israël participent également de ce malaise, sans compter l’éco anxiété et les lourdes interrogations que suscitent le réchauffement climatique et ses conséquences sur le devenir de la planète et de la biodiversité, donc forcément de l’humanité et de notre civilisation. Nous n’ignorons pas non plus les effets des réseaux sociaux sur les jeunes générations. Ces derniers, qui sont au cœur de leur fonctionnement social, peuvent être les être les vecteurs de stigmatisations et des situations de harcèlement dramatiques que l’on connaît. La santé mentale des jeunes est effectivement un enjeu de santé publique publique majeur. La détection et l’accompagnement doivent former un écosystème efficient et justement dimensionné autour de nos jeunes. C’est tout l’enjeu de la prévention. Alors que notre système de soins peine à répondre à l’ampleur des souffrances psychiques et psychologiques, permettez moi de souligner que c’est vrai sur tout le territoire national, mais plus encore dans les zones rurales. J’en profite pour, une fois de plus, enfoncer le clou

La réalité est terrible. Le nombre de médecins formés en France reste largement insuffisant. Le temps médical fourni en moyenne par chaque praticien diminue. La progression de 15

tout objectif d’amélioration de la santé publique est un leurre ou, pis, de la démagogie. Sur le fond, nous souscrivons à l’objectif de mieux détecter les symptômes de dépression, d’anxiété chronique, de bipolarité, de phobies ou encore, parfois dramatiquement, de pensées suicidaires. Le constat est en effet alarmant 40 % des 18 24 ans souffrent de troubles d’anxiété généralisée, un jeune sur cinq connaît des symptômes dépressifs et près de 25 000 jeunes ont tenté de mettre fin à leurs jours. Ce chiffre insupportable nous interpelle. Et je ne parle pas des addictions diverses… Pour ces raisons, le groupe Union Centriste approuve l’objectif d’ériger la santé mentale des jeunes en grande cause nationale. Nous sommes toutefois perplexes sur notre capacité à mettre en pratique et en œuvre cet objectif, faute de moyens suffisants

Les troubles psychiques toucheraient 13 % des enfants et adolescents, soit plus de 1,6 million de personnes. Selon l’étude, les troubles mentaux étaient en 2019 la première cause de perte d’années de vie

Les médecins généralistes doivent davantage être formés en ce sens. Les services de santé scolaire et les psychologues de l’éducation nationale doivent être renforcés de manière significative. Ensuite, le secteur de la pédopsychiatrie doit être soutenu. La Cour des comptes, dans son rapport de mars 2023, rappelait l’intérêt de ces soins, non seulement, pour leur dimension thérapeutique immédiate, mais également pour leur bénéfice préventif en santé à long terme. 48 % des pathologies psychiatriques des adultes commenceraient avant l’âge de 18 ans. Les maladies psychiques représentent un coût économique de 81,3 milliards d’euros pour la France, soit 3,7 % du PIB. Pourtant, la Cour estime les dépenses consacrées à la prise en charge psychiatrique en établissement à seulement 10,4 milliards d’euros, dont 1,8 milliard d’euros pour le secteur infante juvénile. Malheureusement, nous manquons de personnels. Selon l’Ordre des médecins, il y aurait 2 039 pédopsychiatres en France en 2022, soit 34 % de moins qu’en 2010. Cela représente un praticien pour 294 à 392 besoins de prise en charge. La situation ne va pas aller en s’améliorant : 47 % des médecins habilités à exercer en pédopsychiatrie sont âgés de plus de 60 ans. À continuer ainsi, on comptera moins de 1 000 praticiens d’ici à 2035. Des réformes doivent être entreprises pour accroître les effectifs et rendre l’offre des soins accessible. La Cour des comptes en a brossé les grandes lignes ; nous attendons qu’elles soient mises en œuvre. La santé mentale des jeunes nécessite un effort collectif de notre société. Nous partageons les observations et les conclusions des auteurs de ce texte.

À cet égard, le Gouvernement serait bien inspiré de se doter d’un ou d’une secrétaire d’État à la santé mentale, en complément du délégué ministériel, qui devrait être interministériel. Qui d’autre

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, la proposition de résolution de Nathalie Delattre et du RDSE permet d’ouvrir le débat sur un sujet fondamental et préoccupant : la santé mentale des jeunes. Des études récentes confirment, s’il en était besoin, une augmentation significative des troubles de santé mentale, particulièrement chez les jeunes, avec une prévalence croissante de symptômes comme l’insomnie, le stress post traumatique, la dépression ou l’anxiété. C’est une tendance que l’on observe depuis environ cinq ans, mais qui a été accentuée par la pandémie de covid 19, les confinements et les « distanciations sociales », comme nous les appelions, décidés alors. de novembre 2021, l’hôpital Robert Debré lançait un cri d’alarme : les admissions aux urgences pour tentatives de suicide chez les moins de 15 ans avaient augmenté de 300 % en deux ans. La santé mentale doit donc être une priorité absolue, qui se traduit non seulement en paroles et résolutions, mais également par des actions concrètes, des politiques publiques efficaces et des moyens adéquats pour les services de santé. Or, malgré les discours gouvernementaux sur la nécessaire prévention, les moyens alloués aux centres médico sociaux manquent, l’accès aux centres médico psycho pédagogiques est difficile, le remboursement des séances chez les psychologues insuffisant, la médecine scolaire indigente, les équipes médico sociales dans les établissements démunies,

un médecin scolaire. En Seine Maritime, département dont je suis l’élue, quatre postes d’enseignants dans les CMPP de Rouen, du Havre et à Dieppe ont été supprimés l’an passé. Tout cela a des conséquences directes sur la prise en charge de la santé mentale des jeunes et peut avoir des répercussions sur l’ensemble de la société, puisque l’état de santé psychique des enfants et des adolescents est l’un des principaux déterminants de leur santé future. Le dispositif MonParcoursPsy était censé apporter une réponse. Mais moins de 10 % des psychologues s’y sont engagés, faute, notamment, de concertation avec l’ensemble de la profession. Nombre de praticiens nous disent que les 50 millions d’euros investis

en formant des praticiens et en rouvrant des structures et des lits d’hospitalisation. Il est également crucial d’aborder le contexte contribuant à la progression de tels troubles mentaux et comportementaux chez les jeunes. Le caractère inégalitaire de notre système scolaire et la compétition engendrée par Parcoursup, qui va sans doute s’accroître dès le plus jeune âge avec les classes de niveaux annoncées, sont de nature à créer un stress inutile. La précarité – cela a été évoqué – est aussi en cause. Voilà quelques jours, Santé publique France publiait une étude montrant que les enfants vivant sous le seuil de pauvreté sont trois fois plus souvent hospitalisés pour des problèmes psychiatriques. Les étudiants sont confrontés à la précarité, jonglant entre travail et études pour subvenir à leurs besoins, confrontés à la crise du logement, surtout pour ceux qui doivent suivre des études loin de chez eux, et parfois contraints de solliciter l’aide alimentaire. Il est regrettable que vous ayez refusé d’adopter la proposition de loi visant à créer une allocation autonomie L’anxiété s’accroît également en raison des préoccupations croissantes, telles que le dérèglement climatique ou les guerres à nos portes. Je pourrais également évoquer les inquiétudes relatives à l’emploi et à l’avenir, au sens et à ses conditions d’exercice, qui brisent souvent les aspirations de la jeunesse à une vie épanouissante, ou encore les discriminations sociales, de milieu ou de genre. Tout cela nécessite prévention et accompagnement, mais également un environnement et une qualité de vie sains dans les différents espaces sociaux que sont l’école, le travail, la famille et, plus largement, toute la société. Il importe de donner espoir et confiance dans l’avenir et dans la société. Nous sommes profondément convaincus que la santé mentale doit mobiliser l’ensemble de notre société. Nous voterons donc en faveur de la présente proposition de résolution,

Madame la présidente, madame la ministre, chers collègues, chère Nathalie Delattre, la santé mentale des jeunes est une préoccupation croissante dans la société contemporaine. Les jeunes sont confrontés à de nombreux défis et pressions constants, qui peuvent avoir un impact dévastateur sur leur bien être psychologique. Un autre phénomène se développe particulièrement à l’adolescence, période propice à l’expérimentation de comportements à risques : la consommation de substances psychoactives. Aucun adolescent n’est à l’abri et tous les milieux socioéconomiques peuvent être touchés. Les jeunes qui se tournent vers les drogues et les stupéfiants le font souvent pour échapper à leurs problèmes et fuir leur réalité. Mais, au lieu de les aider, de telles substances peuvent avoir des conséquences très graves sur leur santé mentale. Elles créent une addiction extrêmement difficile à surmonter. L’utilisation de drogues peut entraîner des troubles anxieux, des problèmes de comportement, comme l’agressivité. Elle peut également altérer la capacité de concentration, la mémoire et les fonctions cognitives, conduisant à des difficultés scolaires et académiques, ainsi qu’à des problèmes d’apprentissage pouvant aboutir à une déscolarisation. La consommation de stupéfiants chez les jeunes utilisateurs peut avoir des répercussions profondes sur le fonctionnement du cerveau et causer de graves problèmes de santé mentale, notamment la survenue de pathologies, comme la schizophrénie ou la dépression. Récemment, c’est l’usage détourné du protoxyde d’azote, dit gaz hilarant, qui a fait la une de l’actualité. La recrudescence de cet usage chez les jeunes avec des consommations répétées, voire quotidiennes, peut entraîner d’importantes séquelles. Plusieurs cas graves ont d’ailleurs été rapportés au cours des deux dernières années. Nous devons donc nous attaquer aux racines du problème en identifiant le mal être des jeunes qui les pousse à consommer ces stupéfiants pour fuir la réalité et en leur permettant d’être accompagnés par des professionnels de santé compétents.

Il n’y a ni accès direct aux psychologues ni respect du rythme de chacun, et le choix de professionnels est très restreint. Il convient également de mettre en place un véritable dispositif de consultation auprès des psychologues, sans passage préalable par un médecin et sans restriction des motifs de consultation. Les psychologues nous alertent sur l’urgence de faire de la santé mentale des Français, et notamment des jeunes, une cause nationale. Le public concerné mérite une véritable politique publique d’envergure, coconstruite en concertation avec les professionnels de terrain. Madame la ministre, les conditions de travail dans les structures de soin sont tellement difficiles qu’il est extrêmement compliqué de recruter dans certains secteurs. Quelles sont les mesures concrètes envisagées par le Gouvernement pour renforcer les services publics dans le domaine de la santé mentale ? ? Une revalorisation salariale des métiers de soin dans ces structures, et notamment des psychologues, profession peu revalorisée depuis une trentaine d’années, est elle prévue ?

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, la proposition de résolution de Nathalie Delattre invite donc le Gouvernement à ériger la santé mentale des jeunes en grande cause nationale. Elle s’inscrit dans un contexte particulier, marqué à la fois par la crise de la covid 19, qui a provoqué – on le sait – une dégradation importante de la santé mentale des Français, et par la multiplication des travaux sur la question. Après la lutte contre les violences faites aux femmes en 2018 et la promotion de l’activité physique et sportive cette année, il est donc proposé au Gouvernement d’accroître ses efforts en faveur de la santé mentale des plus jeunes par le biais d’un label dont on connaît la portée médiatique : la grande cause nationale. chère Nathalie Delattre, est en effet sans appel. Les jeunes souffrent. Et ils souffrent la plupart du temps en silence. La crise sanitaire de la covid 19, conjuguée à d’autres phénomènes, dont l’éco anxiété, fait qu’ils n’ont jamais été aussi nombreux. Les chiffres sont éloquents : un jeune sur cinq souffrirait de troubles dépressifs. Près de 43 % d’entre eux ont ainsi déclaré en 2021 s’être retrouvés en situation de détresse psychologique. C’est quatorze points de plus que l’année précédant la pandémie de la covid 19 et la tendance ne semble pas vouloir s’inverser. Une étude de Santé publique France a par ailleurs révélé au mois de juin dernier que les enfants n’étaient pas épargnés, puisque 13 % des 6 11 ans présenteraient « au moins un trouble probable de santé mentale Dans ce contexte, le manque de personnel médical, notamment de pédopsychiatres et de médecins scolaires, et de places en milieu médical a des conséquences directes sur la détection et la prise en charge des plus jeunes, avec les effets et les drames que l’on connaît parfois. Face à ce constat alarmant, vous proposez plusieurs pistes pour mieux accompagner ces jeunes : augmentation du nombre de psychologues et de psychiatres disponibles sur l’ensemble du territoire réforme des missions et renforcement des moyens du service de santé scolaire, qui souffre – nous le savons – d’un terrible manque d’attractivité ; soutien aux centres médico psycho pédagogiques et médico psychologiques, psychologiques, etc. Vous suggérez également de mettre en place des campagnes de sensibilisation sur les dispositifs de prévention existants et les offres sanitaires. Car beaucoup a été fait ces dernières années, à mesure que nous prenions, collectivement, conscience de l’ampleur du phénomène et de la tâche à accomplir. de juin 2018, en cohérence avec les objectifs de la stratégie nationale de santé, le Gouvernement a ainsi adopté sa feuille de route de la santé mentale et de la psychiatrie. Organisée autour des trois piliers que sont la prévention, le parcours de soins et l’insertion sociale, celle ci fixait le cap d’une transformation structurelle et systémique du champ de la santé mentale et de la psychiatrie. Le Ségur de la santé et les Assises de la santé mentale et de la psychiatrie sont venus compléter cette feuille de route en 2020 et 2021, la crise de la covid 19 faisant office – il faut le reconnaître – de révélateur. Parmi ces mesures figurent l’organisation d’une communication grand public, l’amplification du déploiement du secourisme en santé mentale ou la création des maisons de l’enfant et de la famille. Citons également la création du dispositif MonParcoursPsy, qui permet à tous de bénéficier du remboursement de huit séances d’accompagnement psychologique par an, le renforcement du réseau des maisons des adolescents, l’augmentation des effectifs des centres médico psychologiques et du nombre de psychologues dans les maisons et les centres de santé. Ces mesures restent pourtant insuffisantes au regard de l’ampleur de la situation et méritent d’être approfondies. C’est là tout l’objet de votre proposition de résolution. En matière de santé mentale, la question des inégalités sociales et de l’accès aux soins est omniprésente. Les territoires d’outre mer ne font pas exception à la règle. C’est par eux que je terminerai. Au mois de novembre dernier, l’Unicef a produit un rapport, remarqué, consacré aux droits de l’enfant dans ces territoires. Les auteurs y constatent « une situation globalement plus défavorable en matière de respect des droits de l’enfant » et soulignent que le défi de la prise en charge de la santé mentale y est particulièrement difficile à relever alors que l’accès aux soins primaires n’est pas toujours assuré. Je pense notamment à la Guyane et à Mayotte, mais le phénomène est évidemment vérifiable dans l’ensemble des territoires ultramarins, qui souffrent, plus que les autres, d’un déficit d’accès aux soins. Je rappellerai pour finir tout l’intérêt que le groupe RDPI porte depuis des années à la question de la santé mentale, en particulier celle des plus jeunes. Il votera évidemment en faveur de cette proposition de résolution.

jeunes adultes, c’est à dire les publics concernés par la présente proposition de résolution, reste dégradée. C’est ce que confirment divers travaux présentés aux Congrès français de psychiatrie. en 2021, la Défenseure des droits appelait à prendre la mesure de cet enjeu. En 2022, l’Unicef a placé la santé mentale des enfants comme l’un des défis majeurs du III millénaire. En 2018 et 2021, cet enjeu majeur de santé publique figurait au cœur de deux feuilles de route du Président de la République sans que ces appels reçoivent de réponses à la hauteur de l’urgence.

; ensuite, le covid 19, qui a durement frappé et déstabilisé les jeunes alors en pleine période de construction personnelle ; enfin, la situation internationale, économique et sociale complexe. Les jeunes sont aujourd’hui dans un étau, tiraillés entre les angoisses de fin du monde et de fin du mois. À l’occasion du Congrès français de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent de 2023, les professionnels ont constaté que 13 % des enfants et adolescents – cela représente 1,6 million de mineurs,

Partout en France, les sonnettes sont tirées par les services de pédopsychiatrie, débordés. Partout, les institutions sont sous l’eau, confrontées à un manque de moyens financiers, humains, bâtimentaires. À l’hôpital, 30 % des postes de psychiatres à l’hôpital public sont vacants, tandis que le temps d’attente pour un rendez vous en centre médico psychologique (CMP) est, en moyenne, de dix huit mois. Les délais de prise en charge s’allongent pour une première consultation, ce qui aggrave les pathologies de manière considérable. J’en viens viens à la prévention et à l’accompagnement des enfants. En l’occurrence, l’offre de soins est également à mille lieues des besoins. Rendez vous compte : alors que l’on assiste à un vrai virage générationnel dans la prise en charge d’enfants de plus en plus jeunes,

une dizaine de départements ne comptent plus aucun pédopsychiatre libéral à ce jour. Le nombre de pédopsychiatres a été divisé par deux entre 2007 et 2016. L’Association nationale des maisons des adolescents alerte sur la situation d’embolie de toutes ces maisons, partout en France. une faculté de médecine sur cinq n’a pas de professeur d’université en pédopsychiatrie. La dégradation de la santé mentale des enfants et des adolescents appelle une réponse rapide et forte, mais les moyens ne sont pas plus au rendez vous à l’hôpital, à l’école ou dans les universités. Si l’école a pris une part prépondérante dans les déclarations du Président de la République du 16 janvier dernier, on compte un médecin pour 15 000 élèves ! Le temps d’un véritable tournant structurel dans l’organisation de la santé à l’école est il arrivé ? La réponse doit être : oui Pourquoi ne pas former la communauté éducative aux premiers gestes de secours en santé mentale ? Un cours spécifique d’éducation à la santé mentale dans les premier et second degrés existe dans certains pays, comme l’Australie, et les écoles accompagnent le développement psychique, ainsi que la gestion des émotions

réclamant une « stratégie nationale ». Il faut poursuivre ce qui a été engagé et développer les bureaux d’aide psychologique universitaires. La santé mentale des jeunes est également une question de territoires. Face à la complexité d’accès aux dispositifs et structures sanitaires et médico sociaux, face à la longueur des délais pour l’accès aux soins,

de protection maternelle et infantile. Dans les villes, les contrats locaux de santé mentale se multiplient depuis leur création, associant les élus locaux, la psychiatrie publique, les usagers et les aidants. Il en existe 260 en France, couvrant environ 20 millions de Français, Français, mais principalement sur les territoires urbains ; seuls 5 % d’entre eux concernent des territoires ruraux. Leurs financements sont disparates. Il ne peut pas y avoir de différences d’accès aux soins selon le territoire. C’était également le sens de l’appel d’élus locaux lors de la 7 journée nationale des conseils locaux de santé mentale.

mondiale de la santé (OMS) comme une maladie à part entière depuis 2018, ce qui nous renvoie à la question des addictions aux écrans, mais aussi aux paris sportifs, aux jeux d’argent. Je rappelle à ce titre l’amendement adopté dans cet hémicycle sur l’initiative de notre groupe pour renforcer la lutte contre ce fléau.

pour rien dans la baisse de la natalité que nous avons constatée. Car dans un monde aux ressources finies, voire un monde parfois perçu comme fini, la jeune génération ne se projette plus avec des enfants, et l’injonction à la natalité ne fonctionnera pas.

présente proposition de résolution soulignent que la précarité est un facteur de dégradation de la santé mentale. Parce que les jeunes d’aujourd’hui construisent la société de demain, ils doivent disposer de ressources pour pouvoir pour pouvoir aborder l’avenir avec sérénité. Notre groupe partage évidemment très largement un tel constat. C’est pour cela que nous avions souscrit à la proposition de loi de nos collègues écologistes

En cette année de jeux Olympiques, je me permets de rappeler la devise de l’olympisme, « Plus vite, plus haut, plus fort », aux allures d’injonction à la performance, ce qui pèse énormément sur les jeunes et leur santé mentale. Une jeunesse qui va mal est l’assurance d’une société qui se dégradera.

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, près de quatre ans après l’épidémie de covid 19, les effets délétères de celle ci sur la santé mentale des Français sont toujours palpables, comme ceux d’une onde de choc. Les enfants et les jeunes font indéniablement partie des catégories les plus fragilisées sur le plan plan psychologique, entre dépression, anxiété chronique, bipolarité, phobies ou pensées suicidaires. Pour eux, il y a clairement eu un avant et un après covid 19 : entre 2019 et 2021, les admissions aux urgences pédiatriques ont augmenté de 40 %, avec une saturation des lits en pédopsychiatrie. La prévalence des troubles psychiques a doublé parmi les 15 24 ans. La part des étudiants en situation de détresse psychologique est passée de 29 % à 43 %. L’impact de la covid 19 et des confinements successifs sur ces publics vulnérables a fait l’objet, dès le printemps 2020, d’alertes par des professionnels de santé, dont la prise en compte par les pouvoirs publics a cependant été tardive. Rappelons que la campagne nationale de prévention n’a été lancée qu’au printemps 2021, soit un an après le début de la pandémie ! La crise sanitaire, par son ampleur inédite, a surtout mis en lumière les difficultés bien connues de notre modèle de prise en charge que sont le manque de lisibilité, les cloisonnements, les disparités territoriales et les inégalités d’accès ou encore le déficit chronique de financement. Il est grand temps d’y prêter toute notre attention, comme le Sénat a d’ailleurs commencé à le faire dès 2021, avec le rapport d’information de nos collègues Victoire Jasmin et Jean Sol, qui contenait de premières propositions concrètes. Il est tout d’abord indispensable de pouvoir détecter les troubles psychiques dès le plus jeune âge. Pour cela, la médecine scolaire doit être confortée, car elle est un outil décisif de prévention et d’orientation des enfants vers un parcours de soins adapté. Les actions de soutien à la parentalité doivent aussi être érigées en priorité, afin d’améliorer l’accompagnement et le repérage précoce des troubles chez l’enfant et l’adolescent. La méconnaissance et, par voie de conséquence, les préjugés qui entourent la santé mentale chez les jeunes retardent l’accès à une prise en charge, voire entraînent un non recours aux soins. La prévention primaire est encore trop sous développée en France, à défaut notamment de statut spécifique pour les métiers qui s’y consacrent ou de structure adaptée. Il est aujourd’hui nécessaire de renforcer le rôle des psychologues, acteurs clés de la prise en charge de premier niveau en santé mentale. La profession s’estime, à raison, mal reconnue et insuffisamment valorisée dans le système de soins. Si la loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 a généralisé la prise en charge par l’assurance maladie des séances réalisées avec un psychologue dès l’âge de 3 ans, les conditions financières restent cependant peu attractives et la condition de prescription médicale peut encore constituer un frein. La psychiatrie est également le parent pauvre de la médecine. Chacun peut imaginer le désarroi dans lequel se trouvent les familles quand on leur annonce qu’il faut attendre parfois jusqu’à deux ans pour obtenir une place dans un centre médico psycho pédagogique, comme c’est le cas chez moi, au CMPP de Gauchy, dans l’Aisne. Il convient aussi de promouvoir de nouveaux métiers en santé facilitant l’orientation des patients dans le système de soins et œuvrant en faveur de la prévention. Je pense en particulier aux infirmiers en pratique avancée, qui peuvent, depuis 2019, obtenir une mention en santé mentale et psychiatrie. Pour faciliter l’accès aux soins des adolescents et des jeunes, qui restent un public très difficile à capter, il faut soutenir la pratique de l’« aller vers », une démarche proactive qui permet d’aller à la rencontre des jeunes, là où ils se trouvent, afin de les sensibiliser et de les orienter vers des professionnels de santé. Dans l’espace numérique, sur les lieux de vie des jeunes ou encore dans la rue pour les mineurs en errance, des initiatives intéressantes méritent d’être encouragées. La médecine universitaire ne doit pas non plus être oubliée, car elle contribue fortement à rassurer et à aider les étudiants en pleine incertitude quant à leur avenir. L’approche de jeune à jeune, de pair à pair, offre aussi une solution de remplacement efficace aux prises en charge classiques. Elle crée un nouveau rapport fondé sur la confiance et la dimension communautaire de l’accompagnement. Mes chers collègues, quand la société ne va pas bien, nos jeunes ne vont pas bien. Se préoccuper de la santé mentale de nos jeunes, c’est se prémunir contre la délinquance de plus tard ; c’est leur donner une chance de s’insérer dans la vie professionnelle.

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, dans la France de 2024, la psychiatrie est anxieuse ; la psychiatrie est troublée ; la psychiatrie est déprimée. Décrite, à juste titre, comme le parent pauvre du système de soins, la psychiatrie médicale dédiée à la santé mentale figure aujourd’hui parmi les spécialités les moins attractives et les moins choisies par les étudiants en médecine. Cette crise de la psychiatrie, qui touche aussi la psychiatrie infanto juvénile, se traduit fatalement par une insuffisante prise en charge de la santé mentale des jeunes. Est il juste d’ériger cette dernière en grande cause nationale ? Oui, cela va sans dire. est ce suffisant ? Non, évidemment ! La dégradation continue de la santé mentale n’est pas spécifique aux jeunes. Mais il faut rappeler, à la suite de Freud et de la plupart des psychiatres, que c’est dans l’enfance et l’adolescence que se construit la psychologie du futur adulte. C’est là que se joue toute la dramaturgie de la vie psychique de l’individu. C’est donc bien en amont de l’âge adulte que les politiques publiques doivent intervenir, non seulement pour les soins somatiques, mais également pour les soins psychiatriques. Or elles en sont bien loin, et les chiffres sont alarmants ! Depuis 2020, en France, la santé mentale des jeunes ne cesse de se dégrader. Toutes les études tirent la sonnette d’alarme. En 2023, le rapport du Haut Conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge alerte sur l’augmentation de la consommation de médicaments psychotropes par les enfants et les adolescents. D’après la Cour des comptes, 1,6 million de mineurs souffrent d’un trouble psychique. L’acuité de ce problème dans ma région, l’Île de France, a même suscité une question d’intérêt majeur, qui débouche sur un vaste programme de recherche. Ainsi, 78 % des jeunes Franciliens déclarent des signes de dépression modérée ou sévère. Et 25 % ont pensé au suicide ! Ce fléau repose sur des causes multifactorielles, amplifiées par la crise sanitaire : délitement de la sphère familiale difficile accès aux soins, accentué par les inégalités sociales ; emprise des réseaux sociaux ; violence croissante et harcèlement scolaire. Tout cela est aggravé par la stigmatisation sociale persistante des maladies mentales, bien mise en évidence par Maria Melchior, spécialisée dans la santé mentale. Il est plus que temps de neutraliser cette évolution ravageuse. Il faut davantage former les professionnels qui travaillent auprès des enfants au repérage de leurs fragilités. De réels moyens doivent être consacrés à la prévention.

Il faut mettre fin au désengagement de l’État en matière de médecine scolaire, qui est laissée à la charge des communes sans les moyens financiers correspondants. L’État doit recruter des médecins et des infirmiers dans les écoles, des assistantes sociales dans les collèges et les lycées et des accompagnants d’élèves en situation de handicap en nombre suffisant au lieu de mutualiser ces professionnels. L’offre de soins médico psychologiques et psychiatriques doit également être renforcée. Il faut en outre mieux lutter contre le harcèlement, en régulant l’usage des réseaux sociaux chez les plus jeunes et en responsabilisant les parents. Enfin, il est impératif de mieux soutenir les familles et de renforcer la fonction parentale. Rappelons le, les territoires où la parentalité est la moins accompagnée sont ceux dans lesquels la santé mentale des adolescents s’est s’est le plus dégradée ; c’est particulièrement le cas des territoires d’outre mer. Le soutien à la politique familiale passe aussi par le développement d’équipes d’intervention à domicile spécialisées en santé mentale, afin d’accompagner les jeunes mères ou encore par l’allongement et la meilleure valorisation du congé parental.

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, nous le savons tous, la pandémie de covid 19, avec ses multiples impacts dans différentes sphères de la vie, a nui à la santé mentale, notamment celle des adolescents et des étudiants

Les recours aux soins d’urgence pour troubles de l’humeur, idées et gestes suicidaires restent en effet à un niveau élevé chez nos jeunes. Ces derniers étaient plus de 20 % à être concernés par la dépression en 2021, contre moins de 12 % en 2017. À cela, s’ajoute le fait que ces jeunes se préoccupent moins de leur santé mentale ou de leur bien être – comme d’ailleurs de leur santé en général – que leurs aînés. Les récentes données recueillies témoignent donc d’une dégradation de leur équilibre psychologique, mais également d’un tabou encore perceptible autour de ces problématiques. Ces résultats avaient conduit Santé publique France à renforcer la surveillance et la mise en œuvre d’actions ciblées pour libérer la parole autour du mal être. Aujourd’hui, un nouvel axe a été abordé, qui consiste à sensibiliser les jeunes aux activités et aux comportements bénéfiques à leur santé mentale. Par ailleurs, chez les 18 24 ans, les principaux freins à la consultation d’un psy sont le coût, la difficulté à se confier, la crainte de ce qu’ils pourraient découvrir sur eux ou encore celle que l’entourage ne l’apprenne.

Promouvoir la santé mentale, prévenir l’apparition de troubles psychiques et lutter contre la stigmatisation sont des enjeux de santé publique sur lesquels nous devons nous engager pleinement pour accompagner les adultes de demain.

La situation de la médecine scolaire est également très altérée, ce qui ne permet pas aux médecins et infirmiers scolaires d’assurer leurs missions d’accueil, de dépistage et de suivi individuel de l’ensemble des enfants qui le demanderaient. Il paraît nécessaire, la Cour des comptes l’indique dans son rapport sur la pédopsychiatrie de mars 2023, d’améliorer l’organisation de l’offre de soins psychiques infanto juvéniles, et de remédier à une gouvernance peu opérationnelle. Certes, le ministère de la santé a manifesté récemment sa volonté de renforcer l’accès à cette offre de soins, avec la feuille de route de la santé mentale. Cependant, ce programme ne se fixe pas d’objectifs clairs, du point vue tant quantitatif que qualitatif ; surtout elle ne prévoit pas de programmation calendaire pour sa mise en œuvre. L’adoption d’objectifs nationaux de santé mentale infanto juvénile associés à un calendrier précis et à des indicateurs permettrait une évaluation de l’organisation des soins de pédopsychiatrie.